L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Après engagement de la procédure accélérée visant à combattre le harcèlement scolaire. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur cette proposition de loi ont été publiés. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances.

Monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer, qui se trouve aujourd'hui à Strasbourg pour un conseil des ministres de l'éducation, de l'Union européenne, je sais qu'il aurait aimé être présent ce matin à vos côtés, la proposition de loi dont nous allons parler aujourd'hui est importante non seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi pour l'ensemble du gouvernement et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être présente pour débattre du bien-être de nos enfants et de nos adolescents sujet qui me tient particulièrement à coeur et qui est aussi à n'en pas douter, au centre de vos préoccupations ce bien-être est indispensable non seulement. à leur épanouissement mais aussi à leur réussite en transmettant aux jeunes générations les valeurs et principes de la République et en leur enseignant, le respect de la dignité de la personne humaine, nous luttons contre toutes les formes de discrimination et préparons nos enfants à mieux vivre ensemble des cités d'éducation. D'éducation des cités éducative pardon ou encore en créant les petits déjeuners gratuits pour les enfants les plus modestes, nous favorisons l'égalité des chances et mettons nos élèves dans les conditions optimales d'apprentissage et de réussite, mais malgré tous nos efforts parfois certains élèves vivent de grandes souffrances, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, victimes de leurs propres camarades mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, le sujet que nous abordons aujourd'hui est grave, faisant appel à nos souvenirs à ces moments de notre scolarité où nous avons été soit victimes soit témoin de harcèlement scolaire qui ont empoisonné la vie d'un enfant à l'âge de l'insouciance, vous avez probablement toutes et tous un nom ou un visage qui vous revient à la mémoire au moment où je vous parle, j'ai une pensée toute particulière pour Dina, qui a mis fin à ses jours à l'âge de 14 ans au mois de novembre dernier et je pense à la souffrance de ses proches et à la douleur de sa mère, Samira Gonthier, avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger à la suite de ce drame. Moqueries, insultes, humiliations raquette bousculade isolement exclusion peuvent être le lot quotidien d'enfants qui subissent les affres d'autres enfants harceleurs, nous ne nous habitueront jamais à ce que des vies d'enfants et d'adolescents soit brisée, parfois de façon irrémédiable par ce véritable fléau du quotidien et nous devons combattre sans relâche le harcèlement à l'école, partout où ils se trouvent et partout où il s'immisce notons par ailleurs que le harcèlement ne s'arrête pas aux portes des écoles parce que souvent les mêmes victimes et les mêmes harceleur se croisent en dehors des établissements scolaires et parfois dans ce monde virtuel. En effet, si les actions menées depuis 2017 ont permis de contenir le harcèlement physique la progression rapide et exponentielle du harcèlement en ligne droite, aujourd'hui nous alerter et nous conduire à redoubler d'efforts, c'est pourquoi nous avons pris de nouvelles mesures fortes dès 2017 nous avons engagé un plan volontariste et ambitieux pour combattre le harcèlement à l'école, autour de 3 grands axes : prévenir intervenir et formé notre action en matière de prévention s'illustre notamment par l'inscription dans la loi qu'aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement, nous avons également évoqué l'interdiction du téléphone portable au collège, le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le Clemi, la collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les plateformes des réseaux sociaux pour notamment améliorer la prévention du cyber harcèlement, nous avons lancé 5 campagnes de prévention telles que Revenge porn rôle des témoins dynamique de groupe, le 1er degré ou encore le cyber harcèlement et je pense aussi au développement des prix non au harcèlement avec le prix annuel contre le cyber harcèlement lancée en 2017 et le prix spécial écoles élémentaires, lancée en 2019. Aucun n'élève ne doit être laissé seul face au harcèlement et c'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un numéro d'écoute accessible aux 30 20 ainsi qu'un numéro dédié à la lutte contre le cyber harcèlement le 30 18 en partenariat avec l'association, il en France dont je tiens ici à saluer le travail, par ailleurs, nous avons amélioré la prise en charge des situations de harcèlement en renforçant la formation initiale et continue des professeurs, nous avons aussi créé le dispositif des élèves ambassadeurs qui permet la sensibilisation entre les pères et nous avons également mis à disposition des ressources et des guides pour les personnels, les élèves et leurs familles, la lutte contre le harcèlement et l'affaire de tous, ce fléau dépasse nos frontières et c'est pourquoi la France a été à l'initiative de la création de la journée mondiale de lutte contre le harcèlement, fixée au 1er jeudi de chaque novembre à la rentrée scolaire 2021 un nouveau cap a été franchi avec la généralisation du programme phare à l'ensemble des établissements et la mise en place du carré régalien dans les rectorats, la mobilisation de la communauté éducative autour de ce programme aura, j'en suis persuadé des effets significatifs sur le climat scolaire le bien-être de nos enfants et impactera positivement les performances de notre système éducatif, la proposition de loi du député et Juan Balanant, que je tiens à saluer pour son travail et sa détermination s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'ici, elle apporte une nouvelle Pierre à l'édifice, notamment en élargissant la base légale du harcèlement scolaire je connais la mobilisation du Sénat sur ce sujet et je veux saluer particulièrement le travail de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement que vous avez réalisé le harcèlement scolaire n'est pas une fatalité, ensemble, nous pouvons l'éradiquer certains pays certains établissements certains professeurs y parviennent tous les jours et ils doivent nous inspirer pour cela il faut sortir d'une logique exclusivement défensive pour passer à l'offensive, nous devons mener une véritable politique du climat scolaire qui promeut l'engagement des élèves, leur sens de l'intérêt général du civisme. Et de l'empathie ces soft, ceux qui sont essentiels la lutte contre le harcèlement impose la mobilisation de chacun et de chacune des membres de la communauté éducative et au-delà de l'ensemble de la société, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je sais que nos échanges seront nourri et constructif, ce matin, sur ces sujets et je vous remercie pour votre mobilisation. La parole est à monsieur Olivier pas cours, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour 10 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission de la culture, madame la rapporteure, chers collègues, ce n'est pas parce que l'on est petit, que l'on a de petits problèmes, rappelait la dernière campagne annuelle de lutte contre le harcèlement scolaire chaque année ce sont entre 800000 et 1 1000000 d'élèves qui en sont victimes, Ce sont autant de parcours scolaire fragilisé d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes en souffrance parfois encore de longues années après la fin de leur scolarité. Le harcèlement peut aller jusqu'à tuer en 2021, une vingtaine de pré-adolescents et d'adolescents est morte victime de harcèlement scolaire parce que le harcèlement scolaire n'est ni une version moderne de la guerre des boutons, ni un bizutage bon enfant parce que ses conséquences peuvent être tragique parce que des solutions existent, il est impératif d'agir pour briser la loi du silence qui nourrit et fortifie ce fléau mortifère. Permettez-moi d'avoir une pensée au nom de la haute assemblée, pour toutes ces victimes et pour leurs familles meurtries par ce mal dont on doit mesurer toute l'étendue et toutes les menaces, certains sont dans les tribunes, j'ai une pensée particulière pour Pierre. Le Sénat s'est penché il y a peu sur ce fléau en 2019 à l'occasion de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, tout d'abord et très récemment, en septembre dernier par la mission d'information sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, je tiens à saluer les travaux de cette mission sénatoriale présidée par Sabine et donc Colette Mélot était rapporteur le constat dressé et précis et les recommandations pragmatiques, ils nous ont permis d'enrichir ce texte sur plusieurs points, en tant que ministre Luc Chatel, il y a une dizaine d'années s'est saisi le 1er cette question et a cherché à mettre en place une réponse institutionnelle pour mettre fin au harcèlement scolaire à sa suite, tous les ministres de l'Éducation nationale ont apporté leur Pierre au rempart à construire face à ce harcèlement scolaire 10 ans se sont désormais écoulé, quel bilan tirez il y a des actions positives qu'il convient de saluer, je pense à la prise de conscience de la part de l'institution scolaire, il ne s'agit pas de chamailleries d'enfants ou encore à la mise en place de numéro d'appel, que ce soit le 30 18 ou le 30 juin je rends hommage à l'engagement des 2 associations en charge de la gestion de ces 2 bouées pour les élèves et leurs familles souvent désemparées et désespérées, en quête d'un interlocuteur et d'une solution, je salue également l'action de toutes les associations engagées dans la prévention du harcèlement scolaire et la prise en charge des victimes et d'cela mais de nombreux points sont perfectibles, la formation des enseignants notamment, seulement 20 % d'entre eux, indique avoir reçu une formation contre le harcèlement scolaire à peine, un enseignant sur 3 se sent suffisamment armés pour repérer des cas de harcèlement et victimaire cela or le harcèlement or le harcèlement scolaire touche tous les milieux et tous les établissements scolaires, tout est prétexte à harcèlement handicap taille vêtements physique parcours scolaire, voire même la couleur du masque, ou encore l'année de naissance, comme l'a montré la campagne hashtag anti-2010 qui a touché les élèves entrant en 6ème à la rentrée 2021, par ailleurs, les numéros d'appel restent souvent mal connue par les enfants et par leur famille, la mission d'information sénatoriale, regrettait d'ailleurs des horaires souvent trop réduit pour leur ouverture, notamment le soir, à le week-end, or c'est justement à ces moments de la journée et de la semaine lorsque l'adolescent et chez lui, seule façon Tél que sévit le plus, le cyber harcèlement c'est également le cas des centres médico- psychologiques dont les délais de prise en charge des victimes de harcèlement s'avèrent encore trop long et les heures d'ouverture de ces structures incompatibles avec une vie scolaire, vous avez déjà été interpellé sur cette question, monsieur le ministre, ça c'était pour Jean-Michel Blanquer en vain pour l'instant, en outre, le programme phare expérimenté en 2019 dans 6 académies et désormais en cours de généralisation illustrent cette ambivalence entre l'existence d'outils et leur méconnaissance par la communauté éducative, selon les chiffres qui ont été transmis lors des auditions, menée sur ce texte 27 % des écoles élémentaires et 43 % des collèges publics étaient engagés dans ce programme à la mi-novembre, dans le canton dont je suis conseiller départemental il y a 2 collèges, l'un a commencé à mettre en place le programme phare, l'autre n'en a pas entendu parler, j'en viens maintenant au texte déposé à l'initiative de notre collègue député Erwan Balanant dont on connaît l'engagement pour le droit à une scolarité sans harcèlement, une question se pose de nouvelles dispositions législatives sont-elles nécessaires pour mieux prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire alors même que le Parlement à légiférer sur le sujet, il y a moins de 2 ans, certes par de nombreux aspects, la portée de ce texte est principalement symbolique, le droit à une scolarité sans harcèlement est déjà inscrit dans le code de l'éducation, il s'agit également d'une liberté fondamentale qui peut faire l'objet d'un référé liberté ce droit s'applique à tous les élèves, qu'ils soient scolarisés dans des des affaiblissements relevant du public comme du privé. Les élèves peuvent déjà être sanctionné pour des faits commis en dehors de l'établissement s'ils ne sont pas dissociable de la qualité d'élèves, il en est de même pour un harcèlement sur internet entre élèves, la circulaire du 17 août 2014 le mentionne explicitement circulaire demande déjà aux établissements de prendre des mesures face au harcèlement scolaire. Néanmoins, ce texte a une portée pédagogique forte, il inscrit par exemple noir sur blanc le fait que ces actes commis en dehors du temps et et du lieu scolaire peuvent relever du harcèlement scolaire ces clarifications sont importantes pour des situations qui concernent majoritairement des mineurs qu'ils soient victimes Arcelor ou témoin les apports de la commission de la culture pour le titre porte sur 4 points : il s'agit, premièrement de conserver la définition d'un harcèlement scolaire limitée au harcèlement entre pairs bien entendu votre discours, on administre la commission souhaite éviter que ce texte jette une suspicion sur l'institution scolaire en légiférant sur un phénomène dont on ne mesure encore ni l'ampleur ni la gravité, nous aurons à en débattre lors de la discussion des articles mais je tiens à le préciser les sanctions pénales et administratives existe un adulte ils sont enseignants, personnels administratifs ou techniques de l'Éducation nationale ou encore assistants d'éducation peut déjà être poursuivi pour des faits de harcèlement commis sur un élève notre droit prévoit d'ailleurs des circonstances aggravantes lorsque le harcèlement est commis sur un mineur de moins de 15 ans, deuxièmement, il nous a semblé essentiel de protéger le rôle et la capacité d'action du réseau des Oeuvres universitaires en sciences, l'Assemblée nationale a créé une nouvelle mission de prévention contre le harcèlement en milieu universitaire, confié au Cnous et aux couches nos collègues députés proposaient de s'appuyer sur les 1600 référent étudiants mis en place dans le contexte de pandémie afin d'accompagner leur père isolées ou en difficulté, or leur financement n'est pas pérenne et nul ne sait s'ils seront maintenues à la fin de l'année universitaire, c'est la raison pour laquelle la commission a supprimé cette disposition, cela me permet de poser la question des moyens humains dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, agir, notamment en matière de prévention du harcèlement nécessite une présence physique de personnes ressource formés à la prise en charge de ce phénomène à l'image de ce qu'ont entrepris les États scandinaves qui se montre exemplaire et précurseur en la matière, c'est tout le le climat scolaire qui doit être engagée et ce au-delà des divers dispositifs et programme clé en main, mis en place par le gouvernement comme l'a rappelé Benjamin Moinard, sociologue spécialiste de l'école, la stabilité des équipes éducatives et leurs modalités de travail sont primordiales pour identifier les problèmes, il y apporter des réponses immédiates. à cet égard, on ne peut négliger les difficultés rencontrées par de nombreux de trop nombreux établissements qui ne dispose pas des moyens humains et des ressources financières nécessaires, un accompagnement efficient des victimes, je pense notamment à la médecine scolaire. Secteurs en grande souffrance et dans les dispositions de cette proposition de loi qu'on sait de le conseil dont le n'apaiseront pas tous les mots. Troisièmement, il a semblé essentiel à la commission de prendre systématiquement en compte le volet cyber du harcèlement scolaire. Le récent rapport d'information de notre collègue Colette Mélot alerter déjà à ce sujet, les réseaux sociaux par leur puissance, leur anonymat leur viralité et la révolution permanente démultiplie les conséquences du phénomène se crée ainsi un continuum de violences entre l'école et la sphère familiale privée sans que les parents et les personnels éducatifs n'en mesure toujours la gravité, notamment faute de savoir-faire technique, il y a désormais ni répit. Ni abri. Brimades et violences ne s'arrête plus aux murs de l'école, l'Hydra maintenant 1000 têtes et son venin s'insinue partout et sans fin. Une prévention et une lutte systématique contre ce nouveau fléau est donc nécessaire et urgente, enfin les témoins, ces petits héros du quotidien, mis en avant par la campagne annuelle de lutte contre le harcèlement scolaire en 2019 les témoins doivent être mieux prises en compte, il joue en effet un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire, la mission d'information sénatoriale a montré avec justesse le harcèlement scolaire se construit très souvent dans une relation triangulaire entre victimes harceleurs et témoin passif agir sur les témoins, c'est casser la dynamique de groupe et faire comprendre à tous que l'effet subi ne sont ni normaux, ni acceptable aussi, nous avons souhaité qu'ils soient systématiquement pris en compte au même titre que les victimes et l'cela de nombreux amendements vont être apportées pour enrichir ce que la commission a déjà la la taxe portée symbolique, je vous propose d'en faire un texte à portée pédagogique garantissant une action à 360 degrés face au harcèlement scolaire et au cyber harcèlement, il doit avoir vocation a rappelé qu'elle ne saurait être menée sans la mobilisation de l'ensemble des acteurs, les personnels intervenant dans les écoles, les collectivités territoriales, le milieu associatif, les acteurs du numérique, les parents, les parents d'élèves et les élèves bien sûr devront y prendre toute leur part, car cette lutte, c'est l'affaire de tous, je vous remercie. La parole est La parole est à Madame Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission des lois, s'est donc saisie pour avis des articles composant le titre 2 de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire qui tente à l'amélioration du traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire et universitaire, il modifie le code pénal, le code de procédure pénale et le code de justice pénale des mineurs, la commission a souhaité garantir la cohérence de notre droit pénal et s'inscrire dans la continuité de travaux de la commission de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement que présidait notre collègue Sabine et dont le rapporteur était Colette Mélot, le rapport de la commission d'information sénatoriale avait notamment souligné le risque lié à la volonté d'inscrire dans le code pénal un délit spécifique de harcèlement scolaire au seul motif d'affirmer un interdit social et de faire primer le symbole sur l'efficacité du droit, la commission des lois a donc adopté un amendement de réécriture de l'article 4 qui crée ce délit spécifique son périmètre pose en effet question il est assorti d'un quantum de peine difficilement Justitia justifiable au regard de l'objectif de prévention et de réinsertion qui prime en matière de justice des mineurs car ce sont principalement des mineurs qui sont auteurs de harcèlement scolaire, il en a néanmoins semblé à la commission des lois, comme les députés ont pu le souligner et à juste titre, que les faits de harcèlement sur survenant dans les établissements d'enseignement doivent être identifiés et faire l'objet d'une sanction renforcée la nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois réintègre donc le harcèlement scolaire au sein du délit général de harcèlement. Donc il constituera une circonstance aggravante, complétant les circonstances aggravantes déjà prévus. Le fait de caractériser les faits de harcèlement survenus dans les établissements d'enseignants comme une circonstance aggravante permettra donc d'éviter que soient sanctionnés différemment des situations pourtant très similaires dans lequel forcément ne se produit pas. Au sein d'Indiens glissements mais entre élèves d'établissements différents et réunit et réunit parfois sur le même site ou dans le bus de ramassage scolaire. Nous avons également souhaité recentrer la caractérisation du harcèlement scolaire sur les faits impliquant les élèves en effet la proposition de loi met sur le même plan les faits de harcèlement entre élèves. Et ce dont l'auteur et membres du personnel de l'établissement, or, si les faits relevant du personnel des établissements d'enseignement doivent être bien évidemment réprimés lorsqu'ils sont constitutifs de harcèlement, il m'apparaît qu'ils ne peuvent être appréhendés de la même manière. La solution adoptée par la commission des lois, vise donc à assurer la cohérence des infractions et des sanctions, tout en renforçant la prise en compte des faits survenant dans les établissements dans saignement, ça nous semble-t-il, une solution équilibrée sur l'article IV prévoyant la possibilité de saisie et de confiscation de téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux conformément au droit existant, la commission des lois a souhaité tirer les conséquences de 2 décisions du Conseil constitutionnel en matière de confiscation des biens ayant servi à commettre un harcèlement et de réquisition des données de connexion. L'absence de dispositions en la matière sera en effet de nature a gravement entravé la conduite des enquêtes, l'article 5 qui modifie le code de procédure pénale pour favoriser l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes de harcèlement dans le cas d'une procédure pénale déjà recommandé mais non explicitement prévu par la loi, a fait l'objet d'un amendement de coordination, l'article 6 modifie le code de justice pénale des mineurs pour préciser que les sages ordonnée par le juge dans le cas de la mise à l'épreuve éducative peuvent comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire clairement, cela relève du domaine réglementaire, il a donc été supprimé, enfin, l'article 7 renforce les obligations pesant sur les fournisseurs d'accès et d'Internet et les hébergeurs en matière de traitement des cas et de signalement aux autorités des faits de harcèlement scolaire, la commission des lois a eu ce débat à de nombreuses reprises et la commission est en effet convaincue que celle des obligations d'obligations prévues au niveau européen, peuvent être efficaces dans cette attente, les obligations qui pèsent sur les opérateurs en la matière et en matière de lutte contre les formes de harcèlement continueront à s'appliquer.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission madame et monsieur les rapporteurs le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement concerne entre 800000 et 1 1000000 d'enfants, c'est-à-dire 6 à 12 % des élèves qui subissent ou ont subi une forme de harcèlement au cours de leur scolarité, chacun d'entre nous doit prendre conscience de cette réalité et mesurer le drame individuel et collectif que le harcèlement représente pour l'école de la République, nous parlons d'enfants et d'adolescents durablement impactés par les menaces, les humiliations ou les violences physiques dont ils font l'objet n'ayant parfois comme solution que la déscolarisation qui les mène peu à peu à un échec scolaire, ces enfants sont doublement victimes, nous avons pu débattre à plusieurs reprises de ce fléau lors du texte pour une école de la confiance, entérinant le droit à une scolarité sans harcèlement ou encore lors du débat à l'issue de la mission d'information sur le même sujet à l'Automne dernier, si le harcèlement scolaire a longtemps été tabou, le sujet fait désormais l'objet d'une véritable prise de conscience de la part des familles, des établissements et des pouvoirs publics pour contrer ce phénomène une mobilisation générale est nécessaire depuis 10 ans une politique publique a été mis en place par les différents gouvernements pur ou lutter contre ce fléau, ces efforts doivent être poursuivis cette année du coeur en éduquant les élèves d'aujourd'hui que nous formerons les citoyens de demain à ce type de cette proposition de loi remet le sujet au centre du débat tout d'abord je salue le travail de la commission de la culture et du rapporteur, Olivier Paccaud, qui se sont attachés à intégrer, à chaque étape du texte, un élément trop absent de la version issue de l'Assemblée nationale, le cyber harcèlement prolongement du harcèlement scolaire amplifiée par l'aspect meute du phénomène via les réseaux sociaux, les tablettes ou les smartphones le cyber harcèlement ne laissent aucun répit aux victimes la précision était donc nécessaire, par ailleurs, notre groupe soutient la nouvelle définition proposée concert consacrant harcèlement entre pairs une définition trop large du harcèlement scolaire incluant notamment les personnels de l'Éducation nationale risquerait d'entraîner trop de dérives sur la création d'un nouveau délit spécifique proposée par l'Assemblée nationale, notre groupe s'inscrit dans la continuité des travaux de la mission d'information sénatoriale sur le sujet et ceux de la rapporteur de la commission des lois, cherche, nous ne sommes pas convaincus de son utilité, cela pourrait même être contreproductif et créer un sentiment de bonne conscience nuisibles à une certaine nécessaire mobilisation générale, ne laissons pas croire que la création d'un nouveau délit suffira à résoudre le problème, si c'était le cas, nous serions déjà pu le régler à partir des textes existants lors de la discussion du texte, nous soutiendrons les amendements de nos collègues, concernant la possibilité pour un enfant harcelé de changer d'établissement, sans tenir compte des limites de la carte scolaire ainsi que se permettant une instruction en famille, ce dispositif permettra aux élèves de limiter au maximum les risques de décrochage scolaire le caractère faiblement normatif des mesures soumises à l'examen du Sénat reflète la difficulté à traiter du sujet du harcèlement scolaire par la loi, je rappelle qu'ils relèvent principalement des projets d'établissement et des protocoles élaborés par l'Éducation nationale au plus près du terrain. Et concernant le cyber harcèlement de la régulation des réseaux sociaux dans la dans la complexité, appelle une réponse au niveau européen, les enseignants sont par ailleurs trop peu formés pour faire face à cette situation, seulement 35 % d'entre eux se sentent armé pour gérer une situation de harcèlement 83 % des enseignants indique n'avoir jamais reçu de formation dédiée à la prévention et à la gestion du harcèlement, ils sont autant à considérer que la lutte contre le harcèlement doit être considérée comme un enjeu de santé publique, enfin la lutte contre ces phénomènes demande des moyens humains, mobilisant l'ensemble de la communauté éducative, je pense aussi à la médecine scolaire, grande absente dans les établissements à tous les niveaux, c'est pourtant grâce aux médecins scolaire et aux psychologues, que l'on pourra aider le harceleur Les harceler et les témoins à parler détecté alerter, informer accompagné ne pourra se faire sans la médecine scolaire. Pour conclure, je souhaite saluer le travail précis de nos rapporteurs Olivier Paccaud et Jacqueline Eustache-Brinio sur ce sujet ainsi que nos collègues de la mission d'information harcèlement scolaire et cyber harcèlement au moment où le groupe Union centriste va voter en faveur de ce texte, nous pensons aux victimes et à leurs familles, ce texte est une première réponse à leurs souffrances pour réussir à enrayer ce fléau, une loi oui mais des moyens sont nécessaires, je pense, notamment, encore à la médecine scolaire angle mort des politiques publiques, je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Fiolet du groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce texte vise à prévenir les faits de harcèlement scolaire et améliorer leur traitement judiciaire ainsi que la prise en charge des victimes. Cette proposition répond à une réalité douloureuse chaque année 700000 élèves sont la cibles d'intimidation d'insultes, d'usurpation d'identité digitale ou encore de menaces en ligne. En 2021 20 enfants et adolescents victimes de harcèlement scolaire se sont suicidés, la dégradation du climat scolaire et de la dignité des élèves harcelés, amplifié par les réseaux sociaux ne peut nous laisser sans réagir. Aussi, nous soutenons les dispositifs prévus par le texte, telle que la consécration du droit à une scolarité sans harcèlement un renforcement des mesures relatives aux préventions de conduites à risques ou encore la formation obligatoire de l'ensemble des professionnels au contact des élèves. Je salue également la volonté de créer une incrimination autonome pour les faits de harcèlement scolaire, il ne s'agit pas d'une surenchère pénale ou d'une discours réponse disproportionnée, il était en réalité question de consolider un interdit social bien que pour l'instant seulement symbolique, l'ajout par la commission du terme de cyber harcèlement dans l'intitulé de ce projet de loi va également dans le bon sens, le harcèlement ne s'arrête pas à la sortie de l'école, devenant pour certains un calvaire sans répit. J'aimerais toutefois revenir sur un acteur qui n'est selon moi pas assez évoqué, c'est le témoin, nous le savons, le harcèlement, hé bien souvent un phénomène de groupe dans lequel peut évoluer une relation triangulaire entre victimes agresseurs moins je suis conscient que chaque individu réagit avec sa sensibilité, son caractère face au harcèlement et que le silence peut éviter d'attirer l'attention de l'agresseur, mais que l'on soit victime ou témoin la démarche reste la même : il faut parler, nous devons encourager la transformation du témoin passif qui devient complice d'une certaine façon, en témoin agissant protégeant c'est en ce sens que je souhaiterais que les formations de prévention des professionnels au contact des élèves se concentre également sur l'identification des témoins. Outre les témoins passifs et agissant que nous avons évoqués, on distingue aussi les témoins actifs, ils ne sont pas les meneurs des l'hymne Annick d'harcèlement il les encourage où y participe, ce sont des collaborateurs dans la triste acceptation du terme : ne fermons pas les yeux à leur égard, la lutte contre le harcèlement doit devenir une responsabilité partagée par tous, je souhaiterais ainsi une révision des sanctions qu'ils encourent ainsi que la création d'une dénomination juridique nier la complexité du harcèlement c'est minimiser la souffrance des victimes et leur protection. Lutter contre le harcèlement scolaire c'est lutter contres la culture de la violence que nous voyons se développer hélas dans tous les domaines, je ne reviendrai pas sur les violences qui vise des enseignants, des élus sur la violence dans les stades et même sur les terrains avec les contestations harcelant des arbitres par les Stars du football qui sont autant de mauvais exemple pour nos enfants et que dire même du harcèlement verbal de certaines interviews, journalistique qui devient la règle à la télévision, c'est pourquoi ce texte malgré quelques fragilités autour du rôle de témoin est un pas de plus vers une scolarité apaisée, le groupe RDSE soutient cette proposition de loi essentielle pour la notion de respect car c'est bien le respect que nous devons affirmer. La parole est à Madame Sabine Van du groupe suaire pour 6 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de commission, madame, monsieur, les rapporteurs, mes chers collègues, je salue l'initiative de cette proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire qui contribuent au renforcement de la nécessaire prise de conscience collective face à ce fléau et à la mobilisation de tous les acteurs, j'y suis d'autant plus sensible que c'est ce que demandait il y a quelques semaines à la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement que j'ai eu l'honneur de présider aux côtés de notre collègue Colette Mélot qui en était la rapporteur nous passons par la loi, soit, et je regrette que le gouvernement n'est pas immédiatement pris la mesure du travail du Sénat et n'est pas jugé utile ou n'est simplement pas souhaité prendre en considération les conclusions de notre mission d'information, nos 35 propositions sont pourtant simples, pragmatiques, immédiatement applicables, pourquoi attendre à les mettre en oeuvre. C'est pourtant possible dans tous les établissements, j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de dire mon incompréhension au ministre Jean-Michel Blanquer dont je regrette l'absence aujourd'hui sur ce sujet, l'ampleur du phénomène du harcèlement et du cyber harcèlement exige pourtant une action rapide, efficace, car 800 1000 à un 1000000 d'élèves subissent une forme de harcèlement ou de cyber harcèlement durant leur scolarité, certains en venant malheureusement à attenter à leurs jours, et j'ai d'ailleurs aujourd'hui une pensée pour leurs proches, c'est insupportable, et cela doit cesser, c'est pourquoi j'accueille positivement l'initiative de cette proposition de loi de notre collègue député Erwan Balanant la plupart des dispositions de cette PPL vont dans le bon sens, même si certaines relève du symbole parmi les dispositions positives, on note la nouvelle place donnée dans le code de l'éducation à la lutte contre le harcèlement scolaire l'extension de la définition du harcèlement scolaire au harcèlement universitaire et au cyber harcèlement l'application des nouvelles dispositions de lutte contre le harcèlement et le cyber harcèlement aux établissements privés ou encore le renforcement de la formation et de la sensibilisation de l'ensemble des personnels entourant les élèves, je suis aussi favorable à la saisine du matériel Tél ordinateur ayant servi au harcèlement pour les besoins de l'instruction et la confiscation de ce matériel au titre de peine complémentaire, la principale divergence de notre groupe vis-à-vis de ce texte, c'était l'article IV et la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire avec des peines applicables particulièrement lourde, sur proposition de la rapporteure au Sénat cet article 4 a été intégralement réécrit en commission, supprimant le délit spécifique de harcèlement scolaire en le transformant Ci-contre circonstance aggravante du délit de harcèlement, cette nouvelle position répond en partie aux prix, aux préoccupations de notre groupe, je veux rappeler que le rapport de la mission d'information sénatoriale n'avait pas souhaité créer un délit spécifique, préférant miser sur une meilleure prévention a-t-elle renforcement des sanctions pénales risquerait de n'être qu'un tigre de papier qui n'aurait que très peu d'effets, d'autres modifications de nos rapporteurs au Sénat suite aux travaux en commissions vont dans le bon sens, comme les amendements visant à la prise en charge des témoins du harcèlement au même titre que les victimes ou les auteurs, c'était d'ailleurs une des préoccupations majeures de notre mission d'information autre modification positive des travaux en commission du Sénat l'extension de l'obligation pour les établissements scolaires et universitaires de lutter non seulement contre le harcèlement scolaire mais aussi contre le cyber-harcèlement avec modification du titre de la proposition de loi, en conséquence, l'extension de l'obligation d'information annuelle des parents aux élèves est aussi approuvé par notre groupe, cela permet de rappeler aux élèves leur droit, c'est de voir ainsi que leurs ressources en cas de harcèlement en tant que témoin ou victime, le travail du Sénat a contribué, dans certains cas les à l'amélioration de cette PPL mais constitue un recul par rapport au texte initial dans d'autres cas, ainsi l'exclusion du harcèlement en provenance des enseignants, du personnel des établissements, même si ce phénomène est très minoritaire, il existe, il ne doit pas être ignoré notre groupe présentera donc un amendement en ce sens à l'article 1er je regrette également la suppression de l'article 3 bis de la PPL en commission au Sénat cet article entendait renforcer les Liens entre les établissements scolaires et les associations de lutte contre le harcèlement scolaire et de soutien aux victimes, nous présenterons un amendement de rétablissement de l'article 3 bis dans une nouvelle rédaction. Par ailleurs, nous souhaitons rétablir par amendement l'article 6 supprimé en commission qui prévoyait des stages de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire dans le cadre de stage de citoyenneté ou de formation civique existant déjà ce dispositif rejoignant une des préoccupations de notre mission d'information, enfin, je veux exprimer mon incompréhension face à la suppression par notre commission de l'article 7 de la proposition de loi cet article prévoyait l'obligation pour les prestataires de services de communication en ligne de concourir à la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire, je trouve qu'il y a une certaine incohérence de la part de nos rapporteurs a d'un côté affirmé vouloir mieux lutter contre le cyber-harcèlement et d'un autre à supprimer cet article 7 pouvons proposeront donc le rétablissement de cet article en demandant de contraindre les hébergeurs et fournisseurs d'accès internet à renforcer leur concours à la lutte contre ce type de harcèlement, j'espère que la présidence française de l'Union européenne sera l'occasion de progresser sur ces enjeux au niveau européen, mais l'actuelle absence de normes européennes contraignantes ne saurait empêcher le législateur français d'anticiper afin de mieux lutter contre un fléau en plein essor qui touche potentiellement tous nos enfants seront très attentifs au sort réservé à noter nos différents amendements, ce qui conditionnera bien sûr notre position finale sur ce texte et je vous remercie de votre attention. La parole est à madame Nadège Havet pour le groupe RDPI. Monsieur le président, madame la ministre madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, Marion, 13 ans, Éva, elle, 11 ans Dina 14 ans, ils ont tous mis fin à leurs jours parce qu'il ne supportait plus les insultes, les menaces, les moqueries, ils sont très ou plutôt trop nombreux à en être victime à en souffrir au cours de leur scolarité, entre les murs ou sur le Net à tous les niveaux du primaire au supérieur, plus de 700000 enfants sont cassés, abîmés par le harcèlement scolaire tous les ans, selon l'association les Papillons ces enfants, ils peuvent être les nôtres nièce nos cousins, nos voisins qui regarderait son enfant se débattre dans ses cauchemars dans ses peurs perdent confiance en lui, perte de confiance en adultes que nous sommes, nous leur devons d'agir, notre action de législateur est nécessaire et c'est pourquoi notre groupe a souhaité inscrire ce texte dans sa niche parlementaire, je salue ici l'engagement remarquable de notre collègue député du Finistère Erwan dont le texte a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mieux prévenir les faits de harcèlement scolaire et la prise en charge des victimes en proposant aux personnels de l'Éducation nationale, une formation continue relative à la prévention à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire créer ensuite un délit autonome de harcèlement scolaire telle est le texte transmis au Sénat, il entend également améliorer le traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire et universitaire, dans son rapport remis au 1er ministre et qui trouve une traduction devant nous aujourd'hui Erwan allons rappeler se chiffrent en moyenne, ce sont 2 à 3 enfants par classe qui sont stigmatisés malmené moqué et violenté dans des établissements publics, privés, avec des conséquences sur le long terme, entraînant des traumatismes profonds et des fragilités durable cette destruction profonde des personnes harcelées, nous l'avons également entendu ici lors de la mission sur le cyber harcèlement menées par nos collègues Colette Mélot et Sabine Van elle face cet état de fait, de nombreuses actions sont nés ces dernières années, la loi pour une école de la confiance consacrent le droit à une scolarité sans harcèlement un numéro de téléphone est disponible des ressources pédagogiques élaborés plusieurs élèves ambassadeur en collège en lycée peuvent être nommés des référents ont été mis en place le travail avec les associations se renforce l'encadrement de l'utilisation des portables dans les établissements scolaires s'inscrit également dans ce cadre d'action, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école est quant à lui, généralisé suite à l'expérimentation menée cette proposition apporte des réponses supplémentaires, notamment sur le cyber harcèlement nous les soutenons, c'est pourquoi nous souhaitons revenir sur les modifications profondes intervenues en commission et nous avons déposé 6 amendements des timbres de rétablissement, nous en discuterons tout à l'heure, la version initiale faut voter de façon transpartisane nous semblent plus efficace, nous y reviendrons lors des discussions à venir mais nous regrettons les reculs suivant l'exclusion des adultes de la faim, une définition du harcèlement scolaire et sa limitation perd la suppression du délit autonome de harcèlement scolaire pour le transformer en circonstance aggravante, de même que l'exclusion de la lutte contre le harcèlement scolaire dans la mission des pour Dina Marion Éva, elle et tous les autres, je souhaite que l'on dise aujourd'hui, comme l'écrit Calogero dans une de ses chansons, plus jamais ça, je vous remercie. La parole est à Madame Colette Mélot du groupe, les indépendants pour 4 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues en France 800000 à un 1000000 d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire : chaque année, ce problème concerne tous les élèves de près ou de loin, créé à l'initiative du groupe, les indépendants, République et Territoires la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement a contribué à identifier les raisons pour lesquelles les actions mises en oeuvre depuis 10 ans en France n'ont pas encore permis d'éradiquer ce fléau, je souhaite pourtant salué le travail de notre collègue Erwan Balanant au moment de l'examen de sa proposition de loi après l'audition d'un grand nombre d'acteurs institutionnels et associatifs, la mission d'information du Sénat n'avait pas fait le choix de l'approche judiciaire que propose Erwan Balanant à travers la création d'un délit autonome de harcèlement scolaire, nous considérons que les outils existants sont suffisants mais méconnu et peu activés sur le terrain, la généralisation du programme phare en septembre 2021 devait permettre d'améliorer la formation et l'information des différents acteurs, en complément, nous avons proposé un certain nombre de dispositions visant à renforcer à unifier la mobilisation de l'ensemble de la société autour de la lutte contre le harcèlement scolaire au 1er rang de ces propositions figurent l'identification de la lutte contre le harcèlement scolaire comme grande cause nationale, afin de faciliter la prise de conscience générale, j'avais quelques réserves quant à la pertinence de l'article IV, identifié comme étant le pilier de cette proposition de loi, cet article a été délégué au fond à la commission des lois, qui a adopté un amendement de réécriture du dispositif, le harcèlement entre élèves de même établissement constitue une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement moral, fidèle aux conclusions du rapport, nous devons agir en priorité sur la prévention des situations de harcèlement pour cela, la formation du personnel des établissements scolaires en incluant les personnels ne dépendant pas de l'Éducation nationale, l'information des élèves et des enseignants et des parents, c'est très important, l'instauration d'un climat de confiance et d'écoute, propice à la libération de la parole sont primordiales, la commission de la culture, a repris dans le cadre de l'article 1er la proposition du rapport visant à délivrer une information annuelle aux élèves sur les risques de harcèlements et de cyber harcèlement le cyber harcèlement prend souvent naissance dans le harcèlement scolaire et vient en plus, hé bien l'amplifier criantes un continuum jusque dans la sphère privée, je salue donc l'initiative de la Commission de l'inclure de façon explicite dans les différents articles afin d'insister sur cette dimension dématérialisé qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, l'article 3 instaure une formation initiale et continue à à la lutte contre le harcèlement scolaire d'un grand nombre de professionnels particulièrement exposés, en revanche, la commission de la culture, a supprimé 2 articles importants, je le déplore l'article 6 vise à créer un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire destiné aux auteurs des faits avérés de harcèlement je suis favorable au rétablissement de cet article qui est issu du rapport d'information sénatorial, l'article 7 oblige les plateformes à se doter d'un dispositif de signalement accessible à tous, il me semble que cette disposition est essentiel si nous voulons combattre efficacement le prolongement du harcèlement scolaire dans la sphère numérique, il appartient à l'ensemble des acteurs d'agir à leur niveau contre cette violence insupportable qui accable des centaines de milliers d'élèves en dépit de ses réserves, je voterai au nom de mon groupe en faveur de cette proposition de loi parce que tous les outils doivent être actionnés afin d'éradiquer un fléau qui peut marquer toute une vie. La parole est à madame Swann du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur, les rapporteurs, mes chers collègues, devant l'urgence devant les drames qui blesse l'enfance devant la tragédie des jeunesses fracturé je voudrais croire que nous partageons tous ici une conviction l'exceptionnel besoin d'agir pour mettre un terme à l'impéritie à l'incapacité collective qui est depuis trop longtemps nous empêchent de mettre en place des mesures concrètes, efficaces et cohérentes afin de lutter contre le fléau du harcèlement scolaire et du cyber harcèlement je voudrais croire que nous partageons tous, ici, une même vision de l'école, délesté de la violence, redevenu ce sanctuaire du savoir, cet espace préservé où se forge la vie d'adulte. Nos enfants sont des être s'sociaux en construction trop faible pour lutter dans une école dont ils ne peuvent s'extraire madame la Ministre, mes chers collègues, réveillons nous ne commettons pas les mêmes erreurs que celles commises envers les femmes harcelées ou victimes de violences, sortons du silence des non-dits et pas sans enfin à l'action, une véritable action. On ne le martèlera jamais assez : chaque année, le harcèlement scolaire fait près d'un 1000000 de victimes, soit 2 à 3 enfants par classe en moyenne 2 à 3 enfants par classe en moyenne, ce phénomène concerne aussi les jeunes enfants, plus d'un élève sur 10 scolarisés en CE2, CM1 et CM2 est victime de ce fléau qui cause près d'un quart de l'absentéisme recensés dans les établissements du 1er degré. Depuis mon arrivée au Sénat je n'avait sans doute jamais éprouvé avec une telle intensité la dimension tragique du mandat de législateur. Mais nous ne sommes plus ici pour constater, nous ne siégeons pas pour déplorer, encore moins pour décrire une réalité que chaque famille, chaque foyer, chaque établissement connaît de près ou de loin et ce texte est l'occasion d'un sursaut. Il ne s'agit pas d'un grand soir, mais de réponse précise à des mots très concret, il ne s'agit pas de posture mais de solutions utiles, alors je vous propose d'agir par voie d'amendement pour garantir aux chefs d'établissement, la stabilité statutaire des assistants d'éducation qu'il recrute et ainsi renforcer ce qui protège nos enfants pour adapter le règlement intérieur à l'évolution du mal que nous combattons y faire figurer le droit à une scolarité sensible et ainsi que les risques des sanctions encourues lorsqu'un élève harcèle un père par voie numérique. Ce règlement, mes chers collègues, est un peu le Code civil de nos établissements, mais ne nous y trompons pas, nous devrons aller plus loin pour créer un choc des responsabilités. Il les 2 acteurs jusqu'ici trop dans le traitement de ce fléau sociétal, les parents en 1er lieu les parents sont les premiers garants du bon usage des outils numériques, il met entre les mains de leurs enfants, il leur appartient de les accompagner dans cet usage et de définir les règles d'utilisation heure de déconnexion durée d'utilisation, présence du téléphone dans la chambre, la nuit, il est du devoir des institutions de rappeler cette responsabilité aux parents avec la création d'un document opposable en cas de conseils de discipline, je pense par exemple à une charte d'engagement civique obligatoirement signé par les parents et les enfants à chaque rentrée scolaire, cette avancée matérialisera ainsi la responsabilité parentale, trop souvent éludée et rendrait tangible : le respect du entre pairs, conditions de la vie citoyenne. Les plateformes en second lieu, c'est bien sûr au plan européen, qu'elles doivent être rappelés à leurs obligations civiques morales et sociétales, car comment comprendre que les réseaux sociaux sur lesquels naviguent et souvent se noie, nos enfants ne se voient imposer aucune responsabilité sociétale, dès lors qu'un jeune et victimes de leurs travers. Cela se pourra on a mon ont le droit communautaire, comme le prévoit le Digital Services Act qu'il vous revient madame la Ministre de voir aboutir au cours de la PFUE et on l'ferme hissant dans le sens que proposez devant nous, la lanceuse d'alerte aux jeunes aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir sur ce texte, nous en avons aussi l'ardent devoir car la politique n'est pas l'affaire de coup d'éclat, mais au contraire de petits pas de jalons sur pardon et progressif, saisissons-nous de cette opportunité non pour allonger encore la panoplie des lois in exécuté mais pour forger enfin les outils qui nous manque, c'est, je crois pouvoir le dire, en leur présence dans cet esprit que nous rapporteurs ont travaillé à ce que l'amélioration collective et tangible de ce texte ne soit pas un vain mot, merci à eux d'avoir prouvé que la constance ne modèrent en rien l'ouverture aux tierces, propositions. Si le Parlement échoué à protéger l'avenir de la nation qu'qui représentent que pourrions-nous dire à cette jeunesse en construction, comment justifier rions, nous notre inaction dans l'éclosion de leur conscience civique. Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas dessus du groupe écologiste pour 4 minutes.

une fois dans lorsque l'arrêté harcèlement classique ayant lieu dans l'enceinte des écoles s'ajoute aujourd'hui le harcèlement en ligne, les victimes sont désormais agressé jusque chez elle, jusque dans leurs chambres, via les réseaux sociaux ou les jeux vidéo 24 heures sur 24 des couloirs de l'école à l'obscurité et au silence d'une chambre d'enfant, le continuum de la violence devient insupportable, les conséquences sont parfois terribles définitive inacceptable les suicides d'enfants, d'adolescents ont jeté un coup de projecteur terribles une lumière crue inévitables sur cette réalité trop longtemps ignoré la société se saisit enfin du sujet, nous nous saisissons enfin du sujet, mais ce fut d'abord le travail inlassable des associations de victimes ou à la mémoire des victimes, un travail d'alerte l'interpellation de sensibilisation, de propositions que nous devons saluer alors que propose la loi tout d'abord la reconnaissance d'un nouveau droit d'un nouveau principe, celui d'une scolarité sans harcèlement. Et pour faire respecter ce principe dans sa version initiale, la création d'un nouveau délit : celui de harcèlement scolaire assorties d'un panel de sanctions très élevé entre 3 et 10 ans d'emprisonnement et de 45 à 150000 euros d'amende selon la gravité, c'est la voie qui a été choisie par les auteurs du texte initial, soutenu par certaines associations concernées et elle peut se comprendre ce délit nouveau permettrait de mieux caractériser les spécificités de ces agressions par les forces de l'ordre et d'attirer encore davantage l'attention de la société des élèves et de la communauté éducative sur ce sujet, la commission des lois a choisi de réunir cet article préférant intégrer le délit de harcèlement scolaire au sein du harcèlement moral dont ils constitueraient une des circonstances aggravantes, allégeant ainsi les sanctions, 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende cette vision ne sommes plus adaptées à la réalité du harcèlement scolaire nous rappelons ici que les agresseurs comme les victimes ses rôles ce sens d'ailleurs parfois sont des mineurs à qui et qu'ils agissent souvent par phénomène de bandes de meute sans excuser les comportements, il nous paraît plus important de travailler à leur détection précoce à leur prévention. Ils ne sont par ailleurs que l'arsenal judiciaire et administratif à notre disposition, s'est largement étoffée ces dernières années, surtout sur les réseaux sociaux, on a ainsi pu voir des individus promptement interpellés puis déférés pour un seul message des cas de dans le cas des des vagues de harcèlement dont a été victime, il a le coeur du problème pour nous n'est pas là, il est dans l'identification, la prévention et la mise en réseau des acteurs, c'est ce que fait en partie la sa proposition de loi en prévoyant des formations de l'ensemble des acteurs de la sphère éducative et en incluant la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les actions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et l'environnement, mais malheureusement, la commission a supprimé notamment la formation obligatoire du tissu associatif, l'inscription de la lutte contre le harcèlement dans l'émission du cross ou encore les stage de responsabilisation, à la vie scolaire aujourd'hui nos efforts nous attend donc désormais se porter sur les moyens alloués, il serait temps de voir si nous voulons nous doter des moyens à la hauteur des principes que nous prétendons défendre. Ne détournons pas le regard d'une grande partie du problème, l'état de la médecine scolaire dans notre pays est un scandale 900 médecins scolaires et 7700 infirmiers et infirmières scolaires pour 12,5 millions d'élèves dans notre pays soit un médecin pour 14000 élèves et un infirmier ou une infirmière pour 1600 élèves une chute de presse de 15 % en 5 ans, c'est un scandale, la pandémie n'a même pas été un déclic le quoi qu'il en coûte, s'est arrêtée à la porte de l'école, voilà des professionnels au contact des élèves qui pourrait identifier les situations à risques engager le dialogue est alerté, mais avec des moyens humains aussi dérisoire, il nous est impossible de leur confier ces missions, plus largement, mes chers collègues, l'école est perméable aux violences du monde des adultes les injonctions et en en en sont les injonctions permanentes et insensées des paroles qui blessent les assignations et discrimination oui lutter contres seulement passe nécessairement par la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité et pour l'émancipation parler du harcèlement des enfants, c'est avant tout parler de l'exemple que notre société donne à ses enfants et en la matière, il nous reste beaucoup à faire, je vous remercie. La parole est à madame Céline Brulin pour le groupe CRCE et pour quatre minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. 6 à 12 % soit environ un 1000000 d'élèves sont victimes de harcèlement au cours de leur scolarité et l'actualité illustrent régulièrement les dramatiques conséquences du harcèlement qui peuvent aller jusqu'au suicide, à l'image de la jeune Dina en novembre dernier, ces chiffres alarmants appellent une mobilisation générale de l'école, mais aussi de l'ensemble de la société, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il a pris ces dernières années un tour nouveau avec le développement des réseaux sociaux et des applications d'échange, de fait, le harcèlement ne s'arrête plus jamais et s'engouffre partout, jusque très tard dans la chambre de ses enfants, il y a donc un nouveau défi à relever pour protéger ces jeunes d'ailleurs, le Sénat ne se trompe pas en ajoutant la mention de cyber harcèlement dans le titre de cette proposition de loi notre amendement à l'article 7 s'inscrit aussi dans cette logique en proposant de renforcer les obligations de service de messagerie instantanée, afin de faciliter le recours au blocage de numéros dans sa version initiale, cette proposition de loi avaient surtout un caractère symbolique important peu aux instruments juridiques existants, à l'inverse, la création d'un délit spécifique initialement prévue à l'article IV était trop déséquilibrée, pas vraiment applicable et pouvait même s'avérer contre-productif au regard de la nécessaire prise de conscience collective sur le sujet, je tiens ici à saluer le travail de cohérence autour de la réponse pénale effectuée par la rapporteur de la commission des lois, ainsi que le rapporteur de notre commission sur ce texte, la définition du harcèlement scolaire sorti de l'Assemblée nationale qui mettait sur le même plan des adultes et des enfants, a été réécrite le délit pénal créé inapplicable au regard de la notion de discernement et disproportionnée dans son quantum de peine a été supprimée sans déresponsabiliser les établissements et les personnels dans la détection, le traitement et le suivi du harcèlement, mais pour prendre en compte les limites de leurs moyens et de leur mission, la proposition de loi vient d'ailleurs renforcer la formation de l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale et des différents acteurs qui doivent être mobilisées face à ce fléau, les enseignants sont déjà sensibilisés dans les vignes spé mais il est nécessaire d'aller plus loin et de renforcer cette formation nous portons d'ailleurs un amendement sur l'article 3, permettant à l'ensemble de la communauté éducative d'y accéder, une des difficultés en matière de harcèlement scolaire, c'est de pouvoir interpréter les signes de repérer l'isolement progressif des victimes et leur permettre de se confier, mais pour cela il faut et vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, plus de moyens, notamment pour la médecine scolaire, les médecins scolaires suivent en moyenne 12500 jeunes des infirmières sont débordées, on le voit, particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire, les assistants d'éducation, tout comme les directeurs d'école, les principaux de collèges et proviseurs de lycées, voient leur mission sans cesse élargi les psychologues scolaires se font de plus en plus rares et, enfin, il est toujours question de départementalisés les infirmières scolaires au sein des PMI, ce qui risquerait de priver la médecine scolaire, d'un peu plus de moyens encore je m'interroge aussi sur cette obsession si vous me permettez l'expression, de vouloir toujours surchargées l'enseignement moral et civique qui ne bénéficient que d'une demi-heure par semaine, ainsi que les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui doivent traiter de sujets d'enjeux toujours plus vaste, on ne peut pas demander à l'école de régler tous les problèmes de notre société et encore moins quand les moyens d'accompagnement ne sont pas au rendez-vous mais ce texte propose une nouvelle étape dans notre engagement collectif contre le harcèlement scolaire c'est pourquoi notre groupe soutiendra ce texte telle qu'issue du travail du Sénat, je vous remercie. La parole à Madame Anne ventes allant du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, devenue une grande cause nationale, le harcèlement scolaire suscite enfin un intérêt à la mesure des souffrances qu'il engendre, il a hélas fallu nombres d'existences brisées pour que ce fléau quitte la rubrique des faits divers pour s'installer dans le débat public, car si certains drames enfin alerter les autorités, ils ne constituent que l'aperçu le plus tragique d'un phénomène qui a des degrés de gravité très diverses gangrène notre école et notre société, si le droit pour les élèves de vivre leur scolarité sans oppression ni anxiété relève de la cause nationale, elle le mérite donc un engagement sincère et massif au delà des effets de manche législatif, ce ne sont en effet pas quelques sentences votées dans cette enceinte qui mettront fin un mal aussi insidieux qu'ancien qui réclame un combat quotidien au sein de chaque classe couloir de collège au cours de récréation, comme l'ont souligné nos rapporteurs ainsi que collecte mélo dans son excellent rapport de septembre 2021, le délit de harcèlement figurent déjà dans notre code pénal, une qualification superfétatoire ne changera donc pas le quotidien des élèves dont l'enfance ou l'adolescence et saccagé, sans compter que la responsabilité pénale étant fixée à 13 ans les peines d'amendes et de prison seront sans effet sur de nombreux cas de harcèlement qui se manifeste dès l'école primaire. Il reste alors le courage de mener ce travail concret minutieux qui ne s'effectue pas avec des déclarations de principe, mais réclame la mobilisation des moyens humains, d'abord en aidant les enseignants à reconnaître le harcèlement en leur dispensant des formations psychosocial ensuite en coordonnant l'ensemble des professionnels les assiettes dans les établissements et en puisant dans les responsabilités de chacun, les compétences utiles pour combattre le harcèlement, il faut ainsi affirmer la place des assistants d'éducation ces AED indispensables à l'harmonie de la vie scolaire et qui pourrait recevoir des missions de veille éducative dans les moments informels que sont les intercours, j'en profite ici pour soutenir la démarche de ma collègue toi de dont l'amendement proposé propose de prolonger les contrats de ses acteurs essentiels, au-delà de ces 6 ans pourquoi se séparer de personnels expérimentés qui connaissent parfaitement le rate le rétablissement et ses difficultés, il convient également de coordonner les actions des conseillers principaux d'éducation avec celle des assistantes sociales, des infirmières scolaires, des psychologues de l'Éducation nationale, ces intervenants travaillent au plus près des élèves, mais encore faut-il, d'une part, renforcer leur synergie, en leur permettant de décloisonner leurs approches et d'autre, Vaud et d'autre part, pourvoir aux postes vacants combien de personnels de santé manque aujourd'hui dans nos établissements, qui devraient pourtant agir pour la prise en charge des élèves, à titre d'exemple, dans mon département de l'Ardèche, le collège Rokia attend son assistante sociale depuis avril 2021 frappé d'interdit le harcèlement le sanctionnant par la loi est nécessaire, mais la menace du code pénal n'est guère dissuasives chez de jeunes enfants et c'est très en amont qu'il faut agir avant même la commission des faits, il faut pour cela former nos jeunes esprits à travers l'enseignement moral et civique afin de connaître et d'accepter les différences, les équipes mobiles de sécurité, pilotées par les rectorats participent à cette sensibilisation mais ce patient travail effectué sur le terrain doit être renforcée et généraliser les sentinelles constitue une initiative intéressante ce dispositif en formant les élèves au repérage des souffrances de leurs camarades leur permet de s'impliquer en rompant avec cette passivité des témoins dont se nourrit le harcèlement cependant cette éducation des enfants à la responsabilité ne doit pas conduire les adultes à se décharger sur le rôle de ces derniers doit demeurer primordiale, à commencer par celui des parents, c'est la raison pour laquelle il m'apparaît fondamental c'est fondamental de les associer très en amont à la lutte contre le harcèlement, l'école a doublement besoin de pour reconnaître les signes avant-coureurs chez une victime et pour transmettre à leurs enfants l'interdit du harcèlement, aucun enfant ne naît ni ne est victime ni bourreau aussi les parents doivent-ils considérés comme des acteurs incontournables de la lutte contre ces dérives, à travers l'examen qui va s'ouvrir, nous allons certainement enrichir ce texte mais aucune loi ne suppléera la volonté politique, donc vous êtes, Madame la Ministre, la dépositaire, donner à nos professeurs aux équipes accompagnantes à la médecine scolaire, les moyens d'accomplir leur voeu le plus cher, voir chaque élève, prendre le chemin de l'école avec sérénité : je vous remercie. La discussion générale est Close, nous passons à la discussion du texte de la commission. à l'article 1er je suis saisi d'une demande de parole de Madame Sabine Draxler du groupe, les républicains. Merci Merci monsieur le président, madame la ministre, aujourd'hui le harcèlement n'épargne plus personne, quelles que soient leurs conditions sociales ou le territoire où il réside rares nos, nos enfants ou nos petits-enfants qui ne seront pas un jour victime témoin ou auteur alors que les zones urbaines et les territoires prioritaires, confronté depuis longtemps à la dimension présidentielle de ce fléau ont pu bénéficier de dispositifs spécifiques pour tenter de le contenir et soutenir ceux qui en sont victimes, les enseignants en milieu rural, dans le 1er degré dans des territoires éloignés de structures médico-psycho- pédagogique ou socio-éducative, non, il faut bien l'avouer, ni la formation ni surtout la disponibilité nécessaire pour faire face seul et bien souvent isolées à ce phénomène. Dans l'article 1er dont nous allons débattre, il est écrit à l'alinéa IV, les établissements d'enseignement scolaire et supérieurs, publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement, prendre des mesures appropriées, c'est bien sûr développer des programmes ad-hoc des guides et des formations, mais c'est aussi pouvoir recourir à un vivier de personnel en mesure d'intervenir régulièrement et rapidement au sein même des écoles, des personnels formés qui pourront mettre en oeuvre en amont des actions de prévention et en avale un suivi personnalisé des élèves et de leurs familles en cas de problème avéré jusqu'à il y a une dizaine d'années, les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté sur la responsabilité des inspecteurs de circonscriptions assurer cette présence dans les écoles rurales facilement mobilisable, notamment en cas de harcèlement, ils étaient un recours précieux de proximité pour les enseignants ou les parents, ces dernières années, de nouveaux paramètres dont le harcèlement complexifie la gestion des classes et le nombre d'élèves et d'enseignants en difficulté à l'école est en nette augmentation, madame la ministre, une fois la loi adoptée, nous comptons vraiment sur vous pour renforcer la présence de personnel spécialisé au sein des circonscriptions, y compris les plus rurales merci. Madame Le Laure Darcos pour une prise de parole. Merci, merci Monsieur le Président, permettez-moi, au moment d'aborder les discussions de des articles de cette proposition de loi de m'exprimer aussi sur ce sujet si grave affirmé qu'un élève a le droit de poursuive sa scolarité sans être harcelé par ses pairs, relève de l'évidence pourtant le harcèlement scolaire est un phénomène qui s'est banalisé depuis plusieurs années et qui prend une ampleur à la fois inédite et inquiétante, avec le développement des réseaux sociaux certes des programmes de prévention sont mis en un demi uvres dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire mais constitue-t-il un rempart suffisamment solide pour circonscrire ce phénomène et dissuader le harceleur, le drame des réseaux sociaux et d'être le reflet des égarements individuel et collectif d'aujourd'hui, les parents et la communauté scolaire, ce sont bien souvent impuissants face à un phénomène qui peut parfois virer au drame, nous l'avons malheureusement constaté récemment la mission d'information sénatoriale sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, a souligné la pertinence d'une information régulière des enfants sur leurs droits et devoirs ou encore l'existence de numéro d'appel en cas de harcèlement, il s'agit d'une nécessité absolue pour ma part, je crois beaucoup à l'attention portée à la victime qui doit pouvoir bénéficier d'un réel soutien psychologique je crois également à la nécessité de prendre en charge les témoins et je tiens ici à saluer les dispositions adoptées à l'initiative de notre collègue rapporteur Olivier Paccaud concernant les témoins de faits du harcèlement qui doivent comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, enfin je ne saurait assez insister sur les vertus de la sanction à l'encontre des élèves harceleurs, elle doit être implacable et doit se traduire par l'exclusion de l'établissement, car je ne peux imaginer un instant que celui qu'on écarte de l'établissement scolaire soit juste l'élève harcelé, bien entendu, le principe de réalité doit nous guider et je soutiens sans réserve la possibilité offerte à un élève dont l'intégrité physique ou morale et menacé de s'inscrire dans un autre établissement en bénéficiant d'une dérogation aux obligations de la carte scolaire ou de changer de mode d'instruction pour l'instruction, en famille, en tout et 4 causes, je forme le voeu que cette proposition de loi favorise le rétablissement d'un climat de bienveillance et de fraternité, dont l'école a bien besoin et j'ai bien entendu une pensée plus qu'émue pour les victimes et leurs familles.

puisqu'il inscrit un droit à la protection contre le harcèlement scolaire au sein du livre au 1er du cote d'éducation et en particulier dans l'Arctique, qui définit les missions. De l'école et des établissements scolaires et donc la lutte. Contre le harcèlement, la protection contre le harcèlement devient une mission et en cela, ce texte est important mais après ce n'est pas parce que l'on ne l'aura écrit dans le code de l'éducation, que la situation sera différente ne nous payons pas de mots, mes chers collègues, ce ne sont pas des injonctions dans le code éducation qui modifient les pratiques qui modifie les les les postures et les positions. ça peut être très clair, a évoqué les moyens qui manquait. On sait que la médecine scolaire que la santé scolaire est en état de on peut ne pas avoir la même position sur les solutions à apporter. Mais on peut être d'accord avec ce constat. Et puis il y a finalement 2 solutions qui peuvent d'ailleurs nous opposer une fois qu'on est d'accord sur le constat. Des moyens supplémentaires, comme l'accident, dit Sabine Dexter mais aussi peut-être aussi de la liberté de la confiance auprès des chefs d'établissement pour leur permettent de régler ces problèmes sans crouler sur de multiples injonctions et de multiples circulaire mais tout simplement en leur faisant confiance pour régler au plus près du terrain c'est problématique et en les formant, pour cela, c'est ainsi qu'on permettra sur ce sujet comme sur bien d'autres, de rénover notre école.

Merci monsieur le président, madame la Nice, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'ouvrir plus largement, comme l'avait fait l'Assemblée nationale, le Champ d'application du harcèlement scolaire et cyber harcèlement, nous souhaitons que toute personne faisant subir une situation de harcèlement à un élève ou un étudiant dans le cadre scolaire ou universitaire puissent être poursuivis, or le texte issu de la commission ne vise désormais que le harcèlement émanant d'élèves ou d'étudiants, nous savons malheureusement que le harcèlement au sein de l'école ou de l'université, peut-être le fait d'adultes, de tels cas sont certes heureusement rarissime, mais existe néanmoins une étude de l'IFOP de mars 2021 réalisé pour l'association Marion Fraisse, la main tendue en fait état, ainsi, selon une étude 3 % des cas de harcèlement scolaire proviendrait d'adultes exerçant au sein de l'établissement, certains de ces cas de harcèlement peuvent avoir les mêmes conséquences dramatiques que ceux en provenance des pères, je citerai ainsi l'exemple de la petite Éva, elle, harceler, notamment par l'un de ses professeurs qui a mis fin à ses jours en juin 2019 elle avait 11 ans, il n'y a donc aucune raison pour que les adultes certes souvent irréprochable exerçant au sein des établissements soient exclues du dispositif, l'argument du rapporteur, selon lequel les arts, les adultes peuvent être sanctionnés ne tient pas puisqu'ils échapperont ainsi aux nouvelles circonstances aggravantes que constitue le harcèlement scolaire notre amendement vise donc à inclure ces adultes exerçant dans les établissements dans le dispositif de l'article 1er qui précise le Champ d'application du droit à la scolarité et aux études sans harcèlement et par conséquence les facteurs constitutifs de circonstance aggravante au délit de harcèlement je vous remercie.

relatif à la définition des du harcèlement scolaire et à la volonté de la Commission, contrairement au texte initial, venus de l'Assemblée nationale de circonscrire le harcèlement scolaire entre pairs, c'est un débat que nous avons déjà eu ici dans cet hémicycle, notamment en 2000 19 au moment de du du vote de la loi sur l'école de la confiance, vous remplacer Madame le Ministre, avantageusement. Jean-Michel Blanquer, je vais pas le faire parler, à votre place, ou à sa place, mais il s'était exprimé à ce sujet, le rapporteur de l'époque sur ce texte, Max Brisson aussi s'en souvient la position ministérielle était clair : le le harcèlement scolaire c'est avant tout entre pairs, cela ne veut surtout pas dire. Que il ne peut pas y avoir malheureusement des cas de harcèlement d'adultes, professeurs, assistants d'éducation, et ça je ne sais jamais envers un élève. Mais ces cas sont prévus par la loi actuelle, ces cas qui sont inexcusables. Sont punis. Pénalement administrativement et si nous avons souhaité circonscrire la problématique du harcèlement scolaire entre pairs, c'est parce que nous ne souhaitons surtout pas, comme l'a dit tout à l'heure dans son nid, une intervention en discussion générale Annick Billon. Risquaient des dérives permettre d'ouvrir entre guillemets de fissurer l'autorité des professeurs jeter la suspicion sur certains professeurs nous avons malheureusement aujourd'hui dans le monde éducatif, certains parents qui refusent, qui critique l'autorité des professeurs et il ne faut pas leur offrir entre guillemets une arme pour. Attaquer les professeurs, alors il ne s'agit en aucun cas d'un blanc-seing entre guillemets pour les adultes qui oeuvrent auprès de de nos enfants, mais l'immense majorité et c'était d'ailleurs très bien dans la la mission que vous présidiez madame l'immense majorité des cas de harcèlement c'est entre pairs. Les très rares cas où un adulte et malheureusement fautifs, ils sont condamnables et condamnées par la loi, donc restons-en là. Avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je vous remercie, monsieur le président, madame la CNET. L'enjeu de cette proposition de loi et de protéger les enfants contre le harcèlement, quel qu'il soit et quelle que soit la personne ayant commis les faits de harcèlement, qu'il s'agisse d'un autre élève ou d'un professionnel qui travaillerait au sein de l'établissement, le gouvernement est favorable au rétablissement de cette mention, ceci étant dit, l'amendement numéro 34 de Madame avec reprend la version 2 du texte de l'Assemblée nationale et il reprend notamment le délit de harcèlement dont nous souhaitons également le rétablissement aussi je vous demande de bien vouloir retirer retirer cet amendement au profit du numéro 34. Vous maintenez. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et une demande de retrait du gouvernement. Quels sont ceux qui sont en Quels sont ceux qui sont contre, ils s'abstiennent, il n'est pas adopté un amendement numéro 34 Madame avait. L'amendement en revenir à la version adoptée en en séance publique à l'Assemblée nationale, nous regrettons tout d'abord, comme notre collègue l'a fait précédemment que les adultes aient été exclus du dispositif par la Commission : le nouveau droit à la scolarité sans harcèlement introduit par la loi pour l'école de la confiance en 2019 doit inclure tous les faits ceux commis par des élèves, des étudiants ou des adultes, il ne s'agit pas pour nous législateur de porter une quelconque suspicion absolument pas, il s'agit seulement de rendre possible une action dans ce cadre, contre des adultes évidemment minoritaire qui adopteraient des comportements il n'ont pas pris inappropriée le harcèlement d'un élève ou étudiant est le plus souvent conçue comme une violence émanant de ses pairs, mais il arrive et des affaires graves sont là pour le rappeler que des adultes présents au sein des établissements aliments voir initie ce phénomène, il s'agit par conséquent de protéger au mieux les victimes en couvrant toutes les situations envisageables de plus, il nous apparaît pertinent de faire figurer la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les missions des centres régionaux des Oeuvres universitaires et scolaires, ce qui a été retiré en commission et nous le regrettons, je vous remercie. Madame avait donc vous souhaitez rétablir le texte telle qu'il nous est arrivé de l'Assemblée nationale, or nous l'avions effectivement réécrit et il y a 2 points sur lesquels il y a, il y a une divergence, le 1er concerne le cyber harcèlement je n'ai pas entendu un seul. Des orateurs en discussion générale ne pas insister sur l'importance du cyber harcèlement qui démultiplie le fléau désormais, moi j'ai utilisé l'expression ni abri ni répit avec le cyber harcèlement malheureusement la la caisse de résonance allez démultiplier, malheureusement dans votre amendement va vous supprimer, vous supprimez ni plus ni moins bon l'alinéa IV le terme de cyber harcèlement à 2 reprises bien alors que pour nous c'est essentiel d'ailleurs, nous avons modifié le type de la proposition de loi en rajoutant le mot cyber harcèlement, deuxièmement, concernant le rôle des que tous ces des trousses, ils ont déjà assez de travail comme ça et donc, il nous semble que leur donner une mission supplémentaire via les 1600 référents qui qui qui ont été nommés et qui bénéficie de moyens pour le budget actuel mais dont on ne sait pas ce qui sera dans le futur, cela ne nous semble pas une une mesure sage, d'où notre volonté de de modifier le texte initial, c'est un avis malheureusement défavorable. L'avis du gouvernement. Merci monsieur le président. que nous légiférons spécifiquement sur le harcèlement scolaire sous toutes ses formes, hé bien la loi doit embrasser toutes les situations possibles, et vous avez évoqué également à la question du cyber harcèlement question que j'ai abordé dans ma prise de parole et je pense que c'est une composante. Complète de du du harcèlement et donc elle est prise en compte en tant que tels, donc par conséquent j'émets un avis favorable. Merci Je suis et très mal à l'aise avec la position du gouvernement et de la majorité présidentielle, je vous demande quel message cela envoie à des fonctionnaires d'État, à des agents de l'État, professeurs et autres fonctions exercées dans les têtes, c'est un petit rond scolaires qui sont des fonctionnaires. Qui appliquent la loi, qui sont soumis à la loi et qui lorsqu'il faute sont soumis à des sanctions. Et avoir des attitudes inappropriées vis-à-vis des enfants. C'est une faute grave pour un professeur qui est déjà sanctionné. Quel message on envoie de considérer que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Que la question de harcèlement entre pairs soit posée et que ce texte soit nécessaire et j'ai dit en discussion de l'article 1er combien c'était un moment important, je le comprends, je le partage, je de soutien mais que l'on dérive vers une suspicion vis-à-vis des agents de l'État, soumis à des règles a des devoirs et des obligations. Et avec une panoplie de sanctions déjà dans les textes, c'est un mauvais message à un moment où la défiance est grande. Entre le ministère et les professeurs de ce pays. Je ne comprends pas, je suis mal à l'aise aussi je soutiens ce que le rapporteur a dit sur le cyber harcèlement, sauf à vouloir reprendre où le texte de l'Assemblée de manière stricte et ne pas considérer que la Haute Assemblée et là aussi, pour enrichir ce texte, je ne peux pas comprendre votre attitude sur le cyber-harcèlement quant aux causes, permettez-moi de dire. Je disais tout à l'heure qu'on se paie de mots on peut multiplier les injonctions, on peut se donner bonne conscience, puis a des réalités, donc on est très loin des réalités, lorsque l'on met une injection supplémentaire de cette nature sur les coups, mais c'est sur le 1er point que je veux dire mon incompréhension, le fait que je sois profondément mal à l'aise vis-à-vis de l'attitude du gouvernement et de la majorité présidentielle sur le sujet. C'est le président madame ministre je je je voudrais insister dans le sens de, de Max Brisson et savoir quelle valeur vous donner encore au statut de la fonction publique c'est l'essentiel est-ce un point sur lequel il faudra que vous exprimiez maintenant, si vous considérez que le statut de la fonction publique est obsolète et qu'il faut lui rajouter des règles spécifiques, je crois qu'on change de régime, madame la ministre, et dans la campagne présidentielle qui vient, nous aurions besoin d'une explication politique forte sur votre volonté de de ce changement de régime par rapport au Cross, je ne comprends pas l'attitude du gouvernement dans cet hémicycle à plusieurs reprises, nous avons souhaité une extension des compétences du cross dans le domaine de la restauration scolaire, notamment par le biais du ticket restaurant, vous l'avez refusé et là vous souhaitez leur donner d'autres d'autres missions pour des des personnes qui sont majeures, ce qui est un ce qui est un problème absolument différent, nous avons besoin maintenant Madame la ministre d'explication sur ce que vous nous proposez, merci monsieur le président.

est aujourd'hui un amplificateur des violences, on ne peut pas se passer de de d'acter dans ce texte, le cyber harcèlement et je remercie à nouveau les rapporteurs dit avoir consacré une partie de leur travail 2ème point sur les trousses alors c'est bien toujours de de donner des nouvelles responsabilités à des organismes mais avec quels moyens on parle de d'harcèlement scolaire on parle de harcèlement comment, avec quels moyens les croûtes vont-ils pouvoir agir contre ce cyber harcèlement c'est impossible, nous sortons d'une audition avec l'art comme l'ARCOM n'est déjà pas en capacité de s'opposer à la divulgation de vidéos pornographiques auprès des mineurs : comment les coûts vont pouvoir combattre le cyber-harcèlement c'est une aberration et concernant le 3ème point sur l'élargissement de la de du harcèlement aux adultes, nous avions hier soir à la demande du président Gérard Larcher une Agora sur l'éducation, hé bien oui, l'éducation, on leur en demande beaucoup, il y a déjà des des règles, il y a déjà des lois en vigueur, qui permettent d'agir donc n'alourdit sont pas le texte ne soit, ne soyons pas plus bavard : les textes existent, ils permettent de condamner ces situations non, nous on à ce qu'il propose la commission les commissions d'ailleurs et je pense qu'on sera dans le vrai, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, évidemment, mesdames et messieurs les sénatrices je je comprends parfaitement les arguments que vous évoquez sur les fêtes que des professeurs puissent être la cible des parents notamment, mais vous l'avez compris, ce n'est pas l'objet de cette loi. Et je rappelle par ailleurs que les enseignants bénéficient déjà aujourd'hui d'une protection fonctionnelle et l'État réagit. Immédiatement, lorsque cela est nécessaire je vous rappelle par ailleurs que le carré régalien qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale permet à la fois de protéger le corps enseignant de prévenir les violences qui peuvent être faites au personnel, il y a également le fait que le le une cellule de lutte est été mis en place au ministère et quelle est là également pour accompagner les enseignants, donc je ne voudrais pas que l'on pense que, aujourd'hui, l'État se décharge de cette responsabilité d'accompagner, de rassurer et de protéger le corps enseignant, mais encore une fois, ça n'est pas l'objet de cette loi, merci. Pardon, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Et un avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent l'amendement n'est pas adopté. Un amendement 20 rectifié madame monsieur Lévy. Oui, monsieur le président, madame la ministre, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le présent amendement permet à la personne harcelée, c'est le désir de pouvoir continuer sereinement sa scolarité ou ses études, le temps que la procédure se met en place et qu'elle aboutisse à l'encontre de la ou des personnes à l'origine du harcèlement par une demande à son rectorat de rattachement, en pratique, on constate que c'est toujours la double peine pour les victimes, non seulement il est harcelé, mais en plus de ça, elle décroche au niveau scolaire, car elle a peur de retourner dans les duels, l'établissement et dire aux chaque jour son ou c'est harceleurs, il faut donc permettre à titre préventif et de façon temporaire de retrouver instamment un établissement d'enseignement dans lequel elle pourra continuer son année d'apprentissage sans risquer de perdre des mois ou une année scolaire, du fait notamment d'une option qui ne serait pas proposé dans un nouvel établissement je vous remercie. Oui, chers Pierre-Antoine Levi, sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais d'autres amendements un peu plus précis que le vôtre, vont arriver, notamment, il y a dans votre ont voté en mousse, parler de procédure, c'est un petit peu vague et je vous demande de le retirer, auquel cas ce serait un avis défavorable, si vous ne lisez pas, il sera satisfait tout à l'heure par d'autres amendements. Du gouvernement. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur Lévy les modalités de traitement des situations de harcèlement permettent d'ores et déjà une réponse rapide et concrète pour lutter contre ce fléau du harcèlement, notamment celles relatives à une prise en charge adaptée des victimes et si le changement d'établissement peut peut constituer une réponse, cette dernière s'apprécie en fonction de la situation de chaque élève, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale en lien avec les maires, s'agissant des élèves du 1er degré dispose d'ores et déjà de toute latitude pour procéder à une nouvelle affectation de l'élève, que cette nouvelle affectation soit dans le secteur dont relève l'enfant ou pas, donc, par conséquent, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Monsieur Lévy vous retirer votre amendement d'accord les retirer. Un amendement 49 rectifié madame Boulet. Merci monsieur le président, mes chers collègues, souvent un chef d'établissement ne prend pas de sanctions au motif que la situation de harcèlement est en cours de traitement par la justice, or, d'une part, même si un comportement n'est pas pénalement répréhensible en raison du manque de preuves suffisantes par exemple, il peut, et c'est souvent le cas avoir enfreint le règlement intérieur de l'établissement scolaire, en outre, le temps de la justice et celui du scolaire n'est pas le même plusieurs années peuvent s'écouler entre le harcèlement subi par l'élève et la réponse pénale, la victime, mais aussi les témoins peuvent alors avoir l'impression que les cas de harcèlement ne sait pas punis dans l'établissement, conformément aux recommandations du rapport d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, cet amendement propose de lutter contre le sentiment d'impunité en distinguant sanctions judiciaires et sanctions scolaires. Madame la sénatrice Céline Boulay-Espéronnier on connaît votre engagement pour la lutte contre le harcèlement scolaire, vous étiez vice-présidente de la mission d'information, néanmoins je je je suis défavorable à votre amendement parce que si vous avez tout à fait raison sur le fait. Il faut décorrélées la sanction pénale de la sanction administrative et que parfois le temps de la justice, comme vous l'avez fort bien dit, est un peu long, dans l'immense majorité des cas, les chefs d'établissement font tout à fait correctement leur travail sanctionne, corrige et protège les élèves victimes de harcèlement, alors peut-être que dans les directives ministérielles et c'est le cas avec le programme phare, il faut insister là-dessus, les formations qui vont être améliorés axés sur cette problématique de harcèlement scolaire pourront insister dessus mais cette amendement me semble jeter un petit peu là un mauvais voile ou une suspicion sur le rôle de certains directeurs ou proviseurs ou principaux de collège et c'est pour cela que j'y suis défavorable. Avis du Gouvernement. Madame la sénatrice Boulay-Espéronnier la procédure disciplinaire est évidemment indépendante de la procédure pénale et ce principe général rappelé à plusieurs reprises par le Conseil d'État. Signifie qu'une sanction disciplinaire peut intervenir quand bien même la juridiction répressive n'a pas encore statué et lorsque le conseil de discipline, estime qu'il n'hésite pas de doute sur la matérialité des faits reprochés à l'élève, il peut, selon sa libre appréciation, décidé de poursuivre la procédure disciplinaire et prononcer une sanction sans attendre l'issue des poursuites pénales et en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits, ou sur le lait leur imputation à l'élève en cause, hé bien l'action disciplinaire peut être suspendue jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcé, le chef d'établissement peut par ailleurs interdire à titre conservatoire l'accès de l'élève à l'établissement, en attendant la réunion du conseil de discipline, par conséquent, quand va. L'amendement est déjà satisfait donc, s'il n'est pas satisfait, ce sera un rejet pour nous. Monsieur Bourgi pour une demande d'explication de vote. Merci monsieur le président, madame la ministre, madame, monsieur le rapporteur, chers collègues j'intervient en appui et en soutien à cet amendement, ce qui vient d'être répondu à notre collègue Boulay-Espéronnier c'est la théorie, je vais vous parler de ce qui se passe dans les établissements scolaires et c'est l'élu local qui siège au conseil d'administration de 8 lycées après avoir siégé au conseil d'administration de plusieurs collèges, dans la majorité des cas, lorsque des faits comme ceux-ci se présente naturellement il y a des suites il y a des conseils de discipline. Mais il arrive aussi que ce soit la stratégie de la défausse, qui se présente et qui s'imposent à la victime. Puisque que vos parents a déposé plainte. On va attendent que la plainte aboutisse, que la justice aboutisse et c'est comme ça que la victime se retrouve isolé et que les agresseurs pensent bénéficier d'un sentiment d'impunité qui n'est plus un sentiment, mais une impunité réelle et effective. Ce que je voulais aussi vous dire ce que parfois des chefs d'établissement, prétendent que si les protagonistes se sont rencontrés et côtoyé dans l'établissement scolaire. La situation de harcèlement a débuté dans l'établissement mais s'est développée à l'extérieur, et notamment sur les réseaux sociaux et dès lors que la situation de harcèlement a dégénéré a dégénéré hors de l'établissement, même si c'est dans l'établissement que les différents protagonistes se rencontrent au quotidien, vous avez des chefs d'établissement qui refusent de prendre leurs responsabilités, pourquoi refuse-t-il de prendre la responsabilité parce qu'ils ont peur que leur établissement soit mal noté par ces magazines qui, chaque année, publie la liste des meilleurs établissements de France, en fonction des taux de réussite au bac, mais aussi en fonction des taux d'incivilité, le nombre de conseils de discipline qui sont convoqués et c'est la raison pour laquelle certains chefs d'établissement refuse de remplir leur rôle lorsqu'une situation de cette nature et portés à leur connaissance et la raison pour laquelle je soutiens votre amendement et je le voterai. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent l'amendement n'est pas adopté que mettre aux voix l'article 1er, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent article 1er est adopté. Un article additionnel après l'article 1er. Un amendement 8 rectifié bis madame bourrin. Merci monsieur le président, pour lutter contre le harcèlement, il est impératif d'en parler, car en parler, c'est ouvrir la voie à la libération de la parole, cet amendement vise donc à mettre en place des mesures concrètes permettant que ce sujet soit régulièrement abordé au sein des établissements avec les élèves, à raison d'une fois par trimestre et ainsi nous assurer que les élèves connaissent les réalités du harcèlement, ces manifestations, et surtout les moyens concrets à leur disposition pour l'empêcher de prospérer. la loi avec l'alinéa 5 de l'article 1er prévoit désormais une séance d'information annuelle. Cela n'empêche pas au cours de l'année, notamment en cours d'éducation morale et civique ou au moment de la journée qui est même européenne du harcèlement qui a lieu au mois de novembre qui a été évoqué tout à l'heure, ça ne veut pas pour ça n'empêche pas d'avoir d'autres moments, pour évoquer cette problématique du harcèlement donc faire obligatoirement dans les programmes qui sont déjà très chargées, 3 séances, ça me semble beaucoup, les enseignants sont libres dans le renseignement de rajouter en cours de 2 séances une fois ou 2 des choses relatives à la problématique du harcèlement si ils la vivent au quotidien l'obligé pour tous les enseignants de France 3 séances annuelles, ça me semble trop.

Ah c'est Madame bourra je je me disais aussi merci, monsieur le rapporteur, je veux vraiment insister sur le fait que la détermination à combattre le harcèlement à enclencher une véritable dynamique dans les athées. Il y a 337 référents académiques et départementaux qui sont les interlocuteurs clés pour les élèves qui sont victimes de harcèlement, le 30 20 et le 30 18 sont les lignes qui sont dédiés à l'écoute et au signalement les ressources sur le site, non au harcèlement existe et de temps forts avec la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école et le prix, non au harcèlement ont été mis en place et, depuis cette rentrée scolaire, le programme français anti-harcèlement phare et généralisé à l'ensemble du territoire national et ce programme est piloté par 213 superviseur au niveau académique, s'ils prennent en charge le traitement des situations au plus près des élèves dans les écoles et les collèges, il y a un volet pédagogique à destination des élèves avec 10 heures d'apprentissage via des supports pédagogiques différence sur l'empathie ou encore le cyber et il y a la mise en place également d'un parcours pédagogique par cycle pour développer les compétences psychosociales ce programme combine différentes actions selon une organisation annuelle, précise, qui prévoit notamment la mise en place d'une équipe ressources et qui permet ainsi aux écoles et aux établissements de mettre en oeuvre de manière effective leur plan de prévention et leur protocole de prise en charge, avec des acteurs formés et des outils adaptés à ces phénomènes et vous l'avez tous ces tous dit extrêmement complexe, donc l'amendement étant déjà satisfait, sinon ce sera un rejet. Madame Billon. Oui, merci Monsieur le Président, juste pour intervenir et et souligné que je partage évidemment, on a l'intention de de de toi notre collègue Antoine lorsqu'elle a présenté cet amendement, je voudrais juste redire que on vote la loi aujourd'hui dans la loi il y a ni obligation de 3 séances par an et par niveau à l'éducation à la sexualité, par exemple, c'est dans la loi depuis des années, ce n'est absolument pas respecté ce n'est absolument et donc bah attention aussi à l'application de la loi ensuite sur la formation des enseignants, en réalité, on est face à un phénomène d'ampleur quand même le harcèlement scolaire et que je, je, je pense que former des enseignants sans trop alourdir leur tâche qui est déjà énorme, mais déformée peut-être à des repérages simple et puis, on arrivera à combattre ce harcèlement scolaire, mes chers collègues, à partir du moment où la médecine scolaire sera réellement présente dans tous les établissements qu'ils seront en capacité d'identifier, de repérer d'accompagner et de lutter contre ce phénomène, donc oui c'est, c'est probablement une intention louable mais attention aussi aux bonnes intentions qui ne sont jamais appliquées ou qui existe déjà, je vous remercie. Moi je comprends les bonnes intentions de tonnes pourra étaient centres bourg que font, je peux même les partager, ce n'est pas sur le fond qu'il y a de mon point de vue difficulté dans une école que très peu scolaire il y a la vie scolaire qui la direction de l'établissement, il y a la santé scolaire dans l'État dont on a déjà parlé qu'il faille, sensibiliser, former. Multiplier les préventions pour lutter contre la le harcèlement et pour protéger les enfants, on est tous d'accord, il y a des efforts à faire, et on peut ici écoutez le ministre ce qu'a dit ne nous dit et puis il y a le temps de la classe, et vous savez, le meilleur moyen d'intégrer dans le temps de la classe des sujets comme celui-là, c'est de travailler sur les programmes et les disciplines ne nous payons pas de mots d'abord toute autre action qui vient perturber le temps d'indiscipline a de conséquences sur l'apprentissage des disciplines une école s'étend en collège ou au lycée, c'est encore et avant tout, un professeur, une salle de classe qui fait des programmes, donc s'il y a des sujets, et c'est un sujet, il faut qu'il soit pris en compte dans le Champ disciplinaire, sinon pour le reste, on est comme le dit Annick Billon, on est dans des c'est injonction. Qui sont des circulaires qui, autrefois, dans des classeurs restent dans le bureau numérique du principal, mais d'un autre, d'autres se traduise pas par des réalités et si on devait comprendre ce qu'est la vie de l'établissement et face à une réelle problématique introduisons là dans ce qui est la réalité d'un établissement une classe un professeur qui enseignent des disciplines et des programmes et ne chargeons pas Alix et le pauvre, code de l'éducation, dont l'obésité va commencer à devenir préoccupante. Madame Mellow. Merci monsieur, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crois que nous sommes tous convaincus d'une chose, il faut prévenir l'effet de de harcèlement, nous sommes tous d'accord là-dessus et, ce faisant, il y a eu ces derniers temps une réelle prise de conscience alors malheureusement ce sont des oedèmes, des événements dramatiques qui ont amené l'opinion à se mobiliser sur le sujet, mais nous avons tous conscience qu'il faut agir contre cette ce ce phénomène de société qu'est le harcèlement scolaire alors comment bon bien, nous y travaillons et nos collègues à l'Assemblée nationale y ont travaillé la PPL est là et nous, nous nous nous nous l'examinons ce matin et la commission des lois, la commission des Lois oui, ainsi que la commission de la culture, se sont vraiment investis sur sur le sujet mais je reprends ce qui vient d'être dire par Annick Billon par Max Brisson, on ne peut pas inscrire tous dans la loi et ce n'est pas un imposant 3 réunions par an, que ça va changer la nature des choses beaucoup d'établissements scolaires et je suis allé dans dans de nombreux établissements scolaires

pour ne pas que c'est ce qui est inscrit dans la loi ne soit pas appliquée. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent l'amendement n'est pas adopté. Un amendement 33 rectifié quater. Madame. Merci monsieur le président, donc, cet amendement vise, au travers du règlement intérieur dont ils doivent avoir connaissance et qu'il signe en début d'année scolaire à rappelé aux représentants légaux et aux élèves les sanctions encourues en matière de cyber harcèlement et ainsi formalisé leurs responsabilités mais je profite. De la présentation de cet amendement pour m'adresser à Madame la ministre expliquait que ce n'est là qu'une première étape parce que le domaine réglementaire étant le mieux à même de concrétiser cet objectif, je vous propose de recevoir cet amendement comme une balise qui a la A, qui est à la fois guidé et à cet à cet égard la création par voie décréta d'un document traitant exclusivement des droits et devoirs de chacun en matière de harcèlement et cyber harcèlement dont la signature par les parents et les élèves le rendre opposable, me semble-t-il de manière indispensable pour créer un véritable choc de responsabilité. Avis de la commission. le code de l'éducation me semble particulièrement pertinent tout à l'heure, je crois que c'est toi justement qui a dit que le règlement intérieur, c'était le code civil de l'établissement scolaire, il est évident que le rôle des parents et clé pour lutter contre le harcèlement et surtout le cyber harcèlement responsabiliser les parents, c'est clés et cet amendement, le permettra, j'y suis très favorable. de du gouvernement. Madame la sénatrice bourrin les sanctions qui sont prises dans le cadre scolaire, ont pour objet de. S'unir aux manquements graves ou répétés aux obligations de l'élève, notamment les atteintes aux personnes, qu'elles soient physiques ou verbales et au bien que ce soit des dégradations ou de la destruction et ces sanctions ont un objectif de réparation et d'éducation au collège et au lycée, elles peuvent conduire à une exclusion temporaire ou définitive de la de de l'enfant et les motifs de sanctions sont d'ailleurs présentes dans le règlement intérieur de l'établissement, qui lui-même est porté à la connaissance il est présenté lors du conseil d'école et du conseil d'administration quand il s'agit d'un collège ou d'un lycée et à l'ensemble des parents d'élèves qui doivent en prendre connaissance, au début de chaque année scolaire et qui doivent le signer, la liste des motifs de sanctions présentées dans le règlement intérieur, notamment ceux concernant les actes de violence physique ou verbale permettent également aujourd'hui de traiter les actes de harcèlement ou de cyber harcèlement et d'autre part, le programme phare dont nous avons déjà parlé qui a été mis en place dans les établissements scolaires permet de donner une information aux parents d'élèves sur les usages que font leur enfants du numérique, notamment sur l'usage des réseaux sociaux, par conséquent, nous pensons que votre amendement est satisfait.

au cours de la mission d'information sénatoriale, nous avons beaucoup insisté sur sur le sujet et je pense que l'amendement de toi ne pourra et nous avons indiqué qu'il fallait qu'il y ait des dans les établissements, chaque année, une inscription : bon, on a, on l'a bien dit dans le le le règlement intérieur, il fallait qu'il y ait sur les tableaux d'affichage dès les les numéros bien placé en fin de vraiment des choses pragmatiques qui peuvent être mises en place tout de suite et je crois que, voilà, ça, l'une d'elles un et savent contribuera encore à faire prendre conscience de de ce sujet et ça et et et les parents de cette façon, seront informés parce que l'information des parents est aussi très importante, tant sur le plan général du du harcèlement que sur le cyber harcèlement et les parents doivent pouvoir intervenir et éduquer leurs leurs si le sont eux- mêmes à l'utilisation des des téléphones portables et et et en général du numérique, je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la Coupe de de la commission qui a été jugé satisfait par Madame la Ministre, donc je considère défavorable. Donc, je vais mettre aux voix, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, l'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article premier bis. Quels sont ceux qui sont pour. Contre ou s'abstiennent l'article premier bis est adopté. Je mets aux voix également l'article 2 quels sont ceux qui sont pour, contre qui s'abstiennent, article 2 est adopté. Un amendement après l'article, un amendement numéro 48 heures, présenté par Madame Cazebonne. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, je vous propose à mon tour une légère modification mais très importante du code de l'éducation à travers son article 452 3 1 et ce afin de lutter encore plus fermement dans nos établissements français à l'étranger contre le frère, le fléau, pardon, du harcèlement je vous propose donc qu'une lutte active deviennent désormais critère d'homologation dans nos établissements, je vous rappelle, à titre d'information, que ça nous avons à travers le monde 553 établissements scolaires à l'étranger. Avis de la commission. Un amendement original mais important parce que le réseau d'éducation française à l'étranger est très important, il ne faut pas l'oublier, donc moi je j'y suis favorable sur le fond, je m'interroge simplement je vais demander l'avis du gouvernement sur la la possibilité de d'évaluer justement cette problématique, donc je demande l'avis du gouvernement. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Cazebonne l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger et la procédure par laquelle. Le ministère en charge de l'éducation, un test et reconnaît que des établissements scolaires situés à l'étranger puisse dispenser un enseignement conforme aux principes au programme et à l'organisation pédagogique du système éducatif français et l'attribution de l'Omo galets de l'homologation s'effectuent en a. D'accord avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et ses principes et ses critères sont appliquées, compte tenu de la législation locale et des accords signés dans les pays d'accueil, l'ajout de ce critère a vocation à s'accompagner d'actions de formation à destination des personnels du réseau de l'enseignement français à l'étranger qui pourront être proposées notamment par l'opérateur public, l'agence pour l'enseignement français en lien avec les formations proposées par le système éducatif français fera ainsi partie des observables pour les corps d'inspection dans le cadre de la procédure d'homologation et de suivi qui est diligentée par le M E N S en lien avec le ministère des Affaires étrangères et son opérateur la EF donc l'application de ce critère devra tenir compte de la la réglementation locale et des accords intergouvernementaux signés par les États d'accueil la règlement stations françaises ne pouvant s'appliquer comme telle à l'étranger ainsi l'ajout explicite du critère de la lutte contre le harcèlement scolaire permet d'inscrire les établissements d'enseignement français à l'étranger, dans la continuité des principes qui prévalent dans le système éducatif français et ainsi d'en incarner les valeurs c'est pourquoi madame la sénatrice, monsieur le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable à cet amendement. En favorable de la commission donc cet amendement, je vais le mettre aux voix qui a reçu 2 avis favorables. Quels sont ceux qui sont cours. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent amendement est adopté. à l'article 3 je suis saisi de deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 35

L'amendement 25 madame Brolin. Merci monsieur le président, j'ai évoqué dans l'intervention générale l'apport très intéressant, me semble-t-il, de la rédaction du Sénat et notamment de cet article 3 qui fait partie des améliorations de ce texte en terme de formation initiale et continue des différents acteurs de la communauté éducative, or dans la liste qui les énumère : il en manque, alors c'est pas pour le plaisir de de rallonger une espèce de liste à la Prévert, c'est que si je prends par exemple, les AESH d'abord il ils demandent régulièrement reconnaissance et qu'on les reconnaisse dans ce texte de loi, ça fait partie je pense de leurs attentes, mais parce qu'on sait aussi que des élèves handicapés sont plus encore que d'autres de potentielles victimes de harcèlement et que dès lors, ce qui les accompagnent, doivent avoir une formation renforcée dans ce domaine-là, je pourrais évoquer les personnels de vie scolaire, qui ont aussi un rôle tout à fait particulier et un lien différent avec les élèves de celui que peuvent avoir les enseignants ou les directions d'établissement qui nécessite là aussi une formation sans doute spécifique et enfin les personnels de direction et je fais écho en cela au débat que nous avons eues précédemment par exemple entre sanction pénale, sanction enfin sanctions judiciaire sanction disciplinaire et qu'il y a aussi dans ce domaine-là à étoffer la formation des des différents acteurs de la communauté éducative, je vous remercie. Avis de la commission. Si Monsieur le Président, alors je dissocie totalement moi les les 2 amendements à l'amendement de Madame avait vise à à rétablir le texte initial venus de l'Assemblée nationale et donc, par exemple, a supprimé la mention des témoins. Je suis totalement défavorable, il faut que les témoins soient pris en considération pour lutter contre le harcèlement pour lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement le rétablissement du texte aussi de l'Assemblée nationale minor ou fait disparaître la notion de cyber harcèlement je suis totalement défavorable à l'inverse, l'amendement de Madame Brulin qui élargit en citant notamment les AESH, hé bien elle a pointé un petit oubli de ma part en tant que rapporteur donc merci madame brûlant et votre amendement j'y suis totalement favorable. Avis du Gouvernement. Madame la sénatrice avait l'article 3 de la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale prévoyait une offre de formation, relative à la prévention à l'identification et à la prise en charge du du harcèlement scolaire cette formation à bord d'heures à toutes les formes que peuvent prendre le harcèlement scolaire y compris le cyber harcèlement et il permettra de construire une culture commune et une réponse globale pour lutter efficacement contre toute forme de harcèlement par conséquent j'émets un avis favorable à votre amendement et en ce qui concerne l'abonnement 25 de madame la sénatrice brûla l'amendement 35 prévoit de réintroduire la rédaction issue de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale cet article se fonde sur l'idée de formation continue proposée à l'échelle de la structure éducative, que ce soit dans les écoles ou les regroupements d'écoles ou les EPL et elle prend donc en compte les AESH qui sont affectés, c'est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement au profit de l'amendement numéro 35. Je vais mettre aux voix l'amendement 35 qui a reçu un avis. Défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour cet amendement, quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent, il n'est pas adopté l'amendement 25 a reçu un avis favorable de la commission et une demande de retrait du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour cet amendement. Quels sont ceux qui sont contre cet amendement est adopté. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 5 rectifier quater Madame Brisson monsieur Brisson, pardon, merci. Si Monsieur le Président, c'est avant, demande que je présente, avec le président Retailleau et de nombreux collègues entend permettre aux parents d'un enfant harcelé de pouvoir le changer d'établissement au cours de l'année ou à la rentrée, sans tenir compte, ai Antoine Lévy des limites imposées par la carte scolaire, lorsque l'enfant est bien impliqué dans son scolaire qu'il a des amis de mon camarade, le changement d'école et peut évidemment être vécu comme un drame et n'est pas forcément dans l'intérêt de faux mais c'est bien cette notion de l'intérêt de l'enfant que nous devons garder à l'esprit lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire car à l'inverse, pour une enfant qui subit les brimades de certains de ses camarades au bout d'en être désocialisés, au point de ne plus vouloir aller en cours, et donc de mettre en péril son avenir une solution doit être trouvée un parent toujours la possibilité d'inscrire un enfant à cet établissement privé, quand même, celui-ci ne serait pas dans son secteur et cela crée une inégalité pour les familles qui ne peuvent pas toutes se permettait ce qui va leur enfant dans un établissement privé, il doit donc être possible de changer leur enfant d'établissement en cours d'année ou à la rentrée, et ceci sans tenir compte des problématiques de la carte scolaire, la rédaction de cet abondement s'appuie sur celle d'une disposition de l'article 49 de la loi, confortant les principes républicains qui permet à une famille de retirer son enfant d'établissements scolaires pour l'inonder l'instruction famille sans interrompre lorsque celle-ci est harcelé à l'école, il s'agit donc de permettre aux mécanismes équivalents pour le changement d'établissement. L'amendement 13 madame Préville. Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement entend permettre aux parents d'un enfant harcelé de le changer d'établissement au cours de l'année ou à la rentrée, sans tenir compte des limites imposées par la carte scolaire, c'est la notion de l'intérêt de l'enfant qui doit nous guider lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire un parent, on l'a déjà dit et a toujours la possibilité d'inscrire un enfant dans un établissement privé, quand bien même celui-ci serait de son secteur et c'est une terrible inégalité pour les familles qui elles ne peuvent pas toujours se permettent d'inscrire leur enfant dans un établissement privé dont les coûts sont parfois importants, ainsi nous devons permettre à des familles de changer leur enfant d'établissement en cours d'année ou à la rentrée, et sans tenir compte de la carte scolaire, je tiens à insister que en matière dans ce de d'harcèlement le maître mot, c'est l'urgence, l'urgence à agir, la rapidité est primordial, faire cesser le harcèlement est un impératif si c'est l'arrêt des souffrances immédiatement, c'est surtout le gage, à long terme de conséquences moindres en réduisant ce qu'on pourrait appeler l'empreinte moral, du harcèlement, la réalité du harcèlement, c'est un traumatisme à vie, la possibilité de changer d'établissement est donc une nécessité tellement d'exemples nous montrent que les parents ayant eu des difficultés à faire changer d'établissement leur enfant ont eu des conséquences délétères pour leur enfant l'école doit rester ce monde et bienveillant pour ce moment si particulier précieux où l'enfant s'ouvre au monde pour apprendre, je vous remercie. L'amendement numéro 23 madame me Pardon. Ben merci Monsieur le Président, cet amendement vise à développer systématiser les solutions d'urgence pour les victimes de harcèlement, selon une note d'information du ministère, de 2015 à collégien sur 5 va changer d'établissement par obligation ou par choix des parents si les causes sont multiples, il faut quand même noter que le climat scolaire et la sécurité ressorti des élèves y sont évoqués néanmoins aujourd'hui une possibilité de changement d'établissement en cas de harcèlement existe cependant cela implique la connaissance par les parents des dispositifs et nous ne pouvons que regretter que cette démarche soit uniquement à leur initiative. Notre amendement propose d'ajouter la mention de la formation à distance par le CNED, c'est un mode de scolarisation, qui n'est pas forcément les plus connus, mais qui peut éviter la phobie scolaire de plus, il nous semble essentiel de faire entrer dans le dispositif, un diagnostic le psy et ce pour 2 raisons : tout d'abord car les enfants en ont très certainement besoin ensuite pour éviter les effets d'aubaine que l'on connaît en matière de carte scolaire merci. Monsieur le président, donc les 2 premiers amendements celui de Max Brisson, cosignée par une cinquantaine de ses collègues, celui d'Angèle Préville, cosignée par elle seule sont strictement identiques, je suis tout à fait favorable pourquoi retirer un enfant de l'école, c'est toujours une défaite de l'école. et ce jamais souhaitable, mais comme l'a dit Madame très ville et comme l'a dit aussi Max il y a des cas où il y a urgence à agir et donc cette dérogation. à la logique de carte scolaire, hé bien il faut effectivement pouvoir y déroger, entre guillemets, Céline Brulin, l'amendement est un petit peu différent, excusez-moi, c'est qui s'exprimer parce que vous rajoutez pour adosser, entre guillemets, c'est cette dérogation, la carte scolaire, la problématique médicale d'un avis médical, or quand on on va de façon précise dans la loi les professionnels qui sont mentionnés et les professionnels de santé au code de 322 1 du code de santé publique, il concerne uniquement la santé mentale et la psychiatrie, or les problématiques de harcèlement scolaire parfois et même souvent aussi ont des faits qui sont physiques, c'est pourquoi je vous demanderai de le retirer ou, à défaut, avis défavorable et avis favorable aux 2 premiers amendements cité. Avis du Gouvernement, madame la ministre. madame Préville j'aimerais rappeler que les modalités de traitement des. Une situation de harcèlement sont permettent déjà aujourd'hui d'apporter une réponse rapide et concrète pour lutter contre ce fléau, notamment celles relatives à une prise en charge adaptée des victimes. Et si le changement d'établissement peut constituer une réponse, cette dernière s'apprécie en fonction de la situation de chaque élève et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale en lien avec les mairies s'agissant des élèves du 1er degré dispose d'ores et déjà de toute latitude pour procéder à une nouvelle affectation de l'élève. Que cette nouvelle affectation soit dans le secteur dont relève l'enfant ou pas d'ailleurs, cet amendement est donc déjà satisfait puisque ce sont les prérogatives du d'Assen concernant l'amendement numéro 23 comme vient de le dire, monsieur le rapporteur, les psychologues de l'Éducation nationale peuvent être saisis à la demande de l'établissement et avec l'accord des parents pour accompagner cette nouvelle inscription et par conséquent le gouvernement est défavorable à cet amendement. Madame Aguirre, pour une demande de parole oui, explications de vote. Oui, nous sommes favorables à la facilitation au changement d'établissement de l'enfant, sans tenir compte des limites de la carte scolaire en cas d'urgence, mais défavorable à la possibilité d'instruire en famille qui revêt pour nous un caractère inégalitaire, je vous remercie.

y compris si c'est pour ce motif-là d'accéder à l'instruction en famille et même nous proposons aussi qu'il puisse bénéficier de l'enseignement à distance, via le CNED, donc ça ne souffre pas débat là-dessus et d'ailleurs ça implique de déroger à la carte scolaire bien évidemment. Cependant, dans notre amendement dont je j'entends qu'il puisse être incomplet puisqu'il n'évoque qu'un diagnostic psy et qu'effectivement il faudrait sans doute élargir ce ce diagnostic, tout en s'appuyant sur la parole de l'enfant, parce que nous sommes absolument convaincus que la parole de l'enfant doit être entrant entendu dans ce genre de situation mais nous nous méfions de faute de garde-fous, je vais le dire comme ça, de la possibilité qui serait ouverte à certaines familles sous couvert, alors je le dis vraiment avec le plus grand respect que je peux avoir pour les victimes, mais sous couvert de harcèlement, d'essayer de déroger à la carte scolaire, donc nous allons maintenir notre amendement tout en en acceptant complètement ce que dit le rapporteur sur ce le fait qu'il soit incomplet en termes de diagnostic pour marquer que il faut quand même que toutes ces dispositions là soient prises dans une perspective de respect de la carte scolaire, je vous remercie. Merci monsieur le président je soutiendrai ces amendements et je regrette juste qu'en tant que maman, que, en fait, ce soit l'enfant harcelé qui souvent doivent changer d'école et ça peut être vie vu comme lui, comme peut-être une punition parce qu'au final il a aussi des amis dans cette école et ben, c'est lui qui doit le plus souvent changer et ce serait vraiment un progrès si ça pouvait être l'enfant harceleurs qui effectivement change d'école. Donc, je vais mettre aux voix. Les 2 premiers amendements qui y sont identiques et qui ont reçu un avis favorable de la commission. Et un avis défavorable du Gouvernement quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contre. Qui s'abstiennent ces des amendements sont adoptés, en revanche, ils sont tombés l'amendement 23 de madame brûle. Je vais mettre aux voix l'article 3 quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contres qui s'abstiennent, l'article 3 est adopté.

Merci, ce président c'était un amendement que je présente, avec le président Retailleau et de nombreux collègues, actuellement, il est encore possible de changer de mode destruction en cours d'année, comme indiqué dans l'article L 131 Thierry steak du code de l'éducation, or l'article 49 de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République qui entre en vigueur à la prochaine rentrée est venu supprimer la possibilité de changement d'instructions en cours d'année, en supprimant les mots, le choix d'instruction il existe aucune raison d'interdire un changement de mode destruction en cours d'année si le mot de nouveau convient mieux à l'enfant, que ce soit pour passer de l'établissement public vers un autre vers une réception privée ou d'un établissement vers l'instruction en famille, il est dangereux de contraindre l'enfant à rester dans un environnement qui ne lui convient pas voir qui peut être nocif pour lui voilà pourquoi opter pour un enfant pour un enfant en danger en cours d'année pour l'instruction en famille doit être une possibilité laissée aux parents qui le qui, tout en le déclarant permettront ainsi de mettre à l'abri leur enfant en danger. L'amendement 42 rectifié bis Madame Boulay-Espéronnier. voire la détresse au coeur de nos débats et de tout favorise enfin favoriser tout ce qu'il est possible de favoriser, pour que l'enfant puisse être extrait s'il est en danger et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, je soutiens et la maman de Max Brisson et. Le mien. Avis de la commission. comme je ai les dit tout à l'heure, retirer un enfant de l'école, c'est toujours une défaite de l'école et c'est jamais souhaitables, on peut changer d'établissement mais il est des cas où effectivement la scolarisation n'est plus possible. Max Brisson l'a très bien dit, dès lors, je donne un avis favorable à cet amendement, mais pour rebondir sur ce que pourrait rétorquer Céline Brulin, oui, effectivement, il ne faut pas instrumentaliser, entre guillemets, la lutte contre le harcèlement à d'autres fins.

de la République prévoit une procédure exceptionnelle afin de permettre aux personnes responsables d'un enfant inscrit dans un établissement scolaire. De solliciter à tout moment l'autorisation d'instruction dans la famille lorsqu'il est établi que son intégrité morale ou physique est menacée et, aujourd'hui, il est déjà donné toute latitude aux Dazed pour modifier l'affectation d'un élève qui serait victime de harcèlement, le gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement. Donc, je vais mettre aux voix, ces 2 amendements identiques qui a reçu un avis favorable de la commission, un avis défavorable du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre ces 2 amendements sont adoptés. Je suis saisie maintenant de trois amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune le cap rectifier quater monsieur Brisson. Merci monsieur le président, c'est à moi de m'en complète le précédent des faits dans le camp où l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée au sein de son établissement scolaire-ci doit avoir le droit d'être de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validations de projets pédagogiques introduites par la loi heures comme pour l'état de santé ou de handicaps des enfants, de pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance afin de permettre à ses enfants un égal accès à l'instruction. Le 14 Madame Préville. doit avoir le droit d'être retiré de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validation d'un projet pédagogique comme pour l'état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance afin de permettre à ses enfants un égal accès à l'instruction. les trois amendements sont similaires, je vais donner un avis favorable, alors je suppose que Madame le ministre, d'Irak, le code de l'éducation permet effectivement de retirer un enfant harcelé de l'école. Sans attendent l'analyse du dossier je pense que c'est ce que vous allez dire, néanmoins il y a toujours la nécessité de présenter un un projet pédagogique pour les parents de montrer leur capacité et cet amendement, il la ligne en fait les les contraintes applicables pour les enfants victimes de harcèlement à de harcèlement scolaire dans leur établissement sur celles qui concernent les enfants victimes de handicaps victime. Victime, c'est peut-être pas le bon mot mais qui ne peuvent pas se rendre à l'école pour cause d'itinérance et aussi d'éloignement géographique, par exemple en zone de montagne, voilà donc il y a une vraie cohérence dans dans dans cet amendement ce triple amendement entre guillemets et j'y suis favorable. l'article L 131 tiré 5 du code de l'éducation prévoit, dans sa version issue de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Qu'une autorisation d'instruction dans la famille peut être délivré pour différents motifs, parmi lesquels l'état de santé de l'enfant ou son handicap, donc l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un enfant peut donc justifier une telle autorisation sur le fondement de ce motif, et par conséquent vos amendements sont satisfaits. Et donc, si vous ne les retirer pas, ce sera un avis de rejet. Je vais mettre aux voix ces ces amendements identiques. Quels sont ceux qui sont pour. Je rappelle que la commission a émis un avis favorable et le gouvernement, une demande de retrait. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Ils s'abstiennent, ils sont adoptés. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 1 Madame Merci monsieur le président, et Madame la Ministre, en fait, cet amendement vise pour certains enfants, qui sont victimes de harcèlement scolaire dont l'intégrité physique ou morale et menacé peut arriver pour un tas de raisons, hein, qu'il n'y a pas de solution alternative, hein, qui est donc une obligation quelque part d'être instruit en famille, l'article 49 de la loi, confortant le respect des principes de la République, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, un stéroïde justement une nouvelle disposition dans le code de l'éducation, stipulant que pour cette déscolarisation d'urgence, elle devait se faire après concertation, alors on a rien contre les les concertations, hein, c'est toujours une très bonne chose de se concerter avec le directeur d'établissement, qui plus est, sauf que les décrets d'la pique la qui vont bientôt sortir en lien avec cette loi, confortant les principes de la République ne dit pas du tout ça, elle précise justement que, il faut une autorisation expresse du directeur d'établissement et comme ça a été très bien dit par monsieur le rapporteur, c'est toujours vécu comme un échec, à juste titre de l'école une déscolarisation vous doutez que mettent la pression sur un directeur d'établissement quant au choix de reconnaître finalement qui a du harcèlement scolaire dans son établissement, c'est le mettent dans une situation très compliquée, ça n'est pas un médecin, ça n'est pas une personne qui est en capacité de dire oui effectivement il harcelé ou non de reposer veut faire reposer cette charge sur ses épaules, c'est une charge malheureusement que certains directeurs d'establishment et j'ai eu de nombreux témoignages ne veulent pas assuré pour ne pas faire de vagues, ne vont pas forcément reconnaître qu'il y a du harcèlement scolaire dans leur établissement, c'est pour ça que cet amendement vise justement à ne pas faire porter cette pression sur les directeurs d'établissements pour la déscolarisation merci. madame Boulay-Espéronnier. Si Monsieur le Président, oui, je vais partir en détail ce que mon collègue vient de dire, mais c'est une forme de de procédure d'urgence, c'est vraiment pour permettre aux familles de bénéficier d'une déscolarisation d'urgence pour l'enfant, quand c'est nécessaire, en urgence, sur justificatif de leur choix, c'est donc une forme de simplification importante, à mon sens, merci. Le de rectifier quater monsieur Brisson. d'après le rapport d'Erwan ou non sur le harcèlement scolaire, les directeurs d'établissement ont tendance à minimiser cela vient d'être dit, les situations de harcèlement, s'il est important de mieux former les Directs établissements à la détection du harcèlement, il est aussi nécessaire de permettre à l'enfant en souffrance d'avoir une solution alternative à la scolarisation dans le cas où son intégrité est menacée de rappelons que la convention était un soldat des droits de l'enfant, signée par la France en 1989 dispose dans son article 12 que l'on donnera notamment à leur fois la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant l'éclaircie de ce droit reste aujourd'hui loin d'être effectif alors que là, que que le code civil portant sur l'autorité parentale, prévoit que les parents à souci d'enfants aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité aussi cet amendement propose d'élargir les critères pouvant mener à une déscolarisation d'urgence en ajoutant le dépôt de plaintes pour faits de harcèlement, il y a des trous, 10 ans, la prise en considération de la parole de l'enfant pour la reconnaissance d'un cas d'harcèlement scolaire. Au numéro 15 Madame Préville. Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, effectivement, comme vient de le souligner parce que c'est le même amendement mon collègue Max Brisson, la convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1989 dispose en son article 12 on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, de même le défenseur des droits, dans son rapport de 19 du 19 novembre 2020 indique de prendre en compte la parole de l'enfant, un droit pour l'enfant un devoir pour l'adulte, rappeler que l'exercice de ce droit reste aujourd'hui loin d'être effectif et nous le constatons et nous voulons l'introduire justement dans cette loi, alors que l'article 371 tirer 1 du Code civil portant sur l'autorité parentale, prévoit que les parents associe l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, la parole du directeur en cela ne suffit pas nécessairement à reconnaître un harcèlement scolaire, celle de l'enfant doit aussi être pris en compte, je vous remercie.

vous l'avez d'ailleurs dit monsieur Chantal c'est toujours préférable et il ne faut pas déresponsabiliser les chefs d'établissement, où vous avez utilisé l'expression veulent faire peser une charge sur. C'est leur métier, ils sont là pour assumer et moi je fais confiance à leur professionnalisme, l'immense majorité font très bien leur travail, donc avis défavorable en ce qui concerne les 2 autres amendements qui sont assez proches, celui de Max Brisson je donnerai un avis favorable, donc c'est important de prendre en compte la parole de l'enfant, madame Préville le souhaite aussi il y a une petite précision supplémentaire qui me paraît très importante dans l'amendement de Max Brisson et de de sa cinquantaine de cosignataires, c'est le fait qu'il appuie sur une plainte. s'est jamais anodin de porter plainte et donc si les parents ont porté plainte, évidemment, l'enfant s'est exprimé, c'est un acte encore plus fort et et je pense que votre amendement, en fait, vous devriez retirer au profit de celui de monsieur. Merci les amendements du sénateur chanterelles et de la sénatrice Boulay-Espéronnier. Permettez-moi de citer précisément ce que dit l'article L 131 5 du code de ceux de l'éducation, dans sa version modifiée par la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, cet article dit lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant et menacé les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnés au 1er alinéa du présent article dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée, les échanges avec l'institution scolaire dans une telle situation, sont tout à fait indispensable et la concertation avec le directeur de l'établissement scolaire est tout à fait nécessaire puisqu'il s'agit là de retirer de l'école, un enfant qui est soumis à à l'obligation scolaire, étant entendu que la scolarisation en établissement reste une priorité et que tout absolument tout doit être fait pour permettre à l'enfant d'en bénéficier, les décrets sur l'instruction dans la famille que le sénateur Chantrel a évoqué tout à l'heure font effectivement actuellement l'objet d'un examen par le Conseil d'État et ils seront probablement prêts d'ici le mois de mai de mai prochain et il prévoit évidemment un dialogue entre les parents et l'établissement et et le 2 le, le directeur de l'établissement, par conséquent, le gouvernement est défavorable à ces deux amendements en ce qui concerne.

de l'article 131 5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 qui traite monsieur le sénateur des situations dans lesquelles l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée et permet aux parents de demander l'instruction dans la concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé est prévue par l'article L 131 tiré 5 et permet de prendre en compte la parole de l'enfant, par ailleurs, le recueil et le traitement de la parole est prévue dans le cadre du programme de lutte contre le harcèlement à l'école et le programme phare élaboré au niveau national par une équipe ressources formé chargée de recueillir la parole des victimes des témoins ainsi que des agresseurs et enfin, comme cela a été dit précédemment, il est déjà donné toute latitude aux dizaines pour modifier l'affectation d'un élève lorsqu'il est victime de harcèlement par conséquent ces amendements sont déjà satisfaits. différemment ces différents amendements, les 2 premiers qui sont identiques ont reçu des avis défavorables et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Contre qui s'abstiennent, donc ils ne sont pas adoptés. L'amendement de monsieur Brisson a reçu un avis favorable de la commission. Et jugé satisfait par le gouvernement, donc défavorable. Quels sont ceux qui sont pour.

Un amendement numéro 28 présenté par Madame brûle. Merci monsieur le président, cet amendement vise à compléter en quelque sorte les objectifs assignés aux visites médicales obligatoires à l'école, qui aujourd'hui se donne l'objectif de détecter les cas de maltraitance et nous proposons d'y ajouté qu'une attention soit portée aux cas de harcèlement d'abord, parce que ces personnels, par définition, on évoquait tout à l'heure les les possibles atteintes à l'intégrité physique de certains enfants victimes de harcèlement, ces personnels de santé sont particulièrement compétent pour les déceler, ils sont aussi compétents pour déceler des signaux qu'on pourrait qualifier de plus faible et donc agir en matière de détection. Et il nous. Donc ça pourrait utilement compléter les dispositifs existants, alors évidemment je devance d'autres amendements et d'autres prises de parole, vraisemblablement, cela nécessite des effectifs de santé scolaire des médecins en particulier et c'est effectivement un enjeu également merci. Bon cher Max Brisson va encore rendre plus obèses le le code de l'éducation, mais je suis totalement favorable à cette proposition pertinente de Céline Brulin, ça nous donne aussi donc que que la détection du harcèlement scolaire fasse l'objet des en partie des visites médicales scolaires, c'est une bonne chose, ça me permet aussi d'évoquer et beaucoup d'entre vous, Thomas dessus Annick Billon Anne talons et Céline Brulin, long, long évoqué lors de leur direction discussion générale il y a la problématique des moyens et notamment de la médecine scolaire, on peut parler aussi des psychiatres à l'école, il y a un vrai problème là-dessus, et alors ce n'est pas l'objet de la loi, mais si on veut être efficace, il faudra évidemment donner plus de moyens, avis très favorable à cet amendement. Avis de du gouvernement. Madame la sénatrice brûla les dispositions prises à l'article L. 542 tiré 2 du code de l'éducation concerne la prévention et la détention, la détection de l'enfance maltraitée. Et à ce titre, les situations de maltraitance qui peuvent être vécues par un enfant, qu'elle soit intra-familial ou scolaire sont évidemment pris en compte par la médecine scolaire et font l'objet d'une attention toute particulière, il n'est donc pas souhaitable de dresser une liste des des situations de maltraitance au risque de, de, d'en éviter ou dans dans nos maîtres quelques-unes et notre avis sera donc défavorable. J'trouvera cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contre, qui s'abstiennent, l'amendement est adopté un amendement numéro 26 heures présenté par Madame brûle. Merci cet cet amendement pardon, prévoit la création d'un rapport sur la prise en charge par la Sécurité sociale, des frais de consultation et de soins engagés pour le suivi d'enfants victimes de harcèlement, on sait que c'est effectivement une manière de soigner, de réparer, si c'est possible, ces enfants victimes mais il nous faut savoir. Notamment parce que un élément assez positif est venu ces derniers temps avec la création du chèque psy, comment sont-ils utilisés ces outils et s'il n'y a pas matière éventuellement à les développer, je crois que par enfin à travers toutes nos interventions nous saluons les mesures qui sont contenues dans ce texte, mais aussi la nécessité d'aller plus loin pour que ce texte ne reste pas en quelque sorte, je vais le dire de manière peut-être un peu maladroite mais seulement nous donner un peu bonne conscience mais vraiment qu'on se dote d'outils très pertinent et performant et je crois que ce rapport nous permettrait de voir à l'avenir, vers quel développement il faudrait travailler pour venir vraiment en aide aux enfants victimes de harcèlement. Avis de la commission. Mais ce sera un avis de sagesse, un avis de sagesse parce que la tradition du Sénat ce n'est pas d'accepter les rapports mais c'est vrai que là on est dans un contexte très particulier et il y a eu la la création l'année dernière, d'une prise en charge psychologique d'un d'un chèque psy dans le cas du confinement, alors quel bilan tirez, bon il y a, il y a beaucoup de questions à se poser et cette ce rapport pourrait être très utile, donc je j'émets un avis de sagesse. Avis du gouvernement. Madame la sénatrice brûlant, vous avez raison de dire que le harcèlement à l'école affecte de manière plus ou moins graves. La santé psychique des des enfants qui peuvent nécessiter une orientation soit vers la prise en charge psychologique soit une prise en charge psychiatrique en fonction des besoins et les assises de la santé mentale et de la psychiatrie que vous avez évoqué tout à l'heure qui ont eu lieu les 27 et 28 septembre dernier ont été l'occasion d'annonces très forte en ce sens, tout d'abord, il existe de nombreuses structures spécialisées aujourd'hui qui propose un accueil et et ou une prise en charge des victimes de harcèlement, les établissements publics tels que les maisons des adolescents ou les centres médico-psychologique, un fantoche juvénile offre un accompagnement psychologique et psychiatrique, lorsque cela est nécessaire, l'objectif pour nous est d'atteindre un ratio d'une maison des adolescents par département en 2000 22 et en 2000 22 et 400 ETPT viendront renforcer les CMP un fantoche juvénile d'ici 2024 il y a également une prise en charge par les psychologues en ville qui est maintenant possible et enfin l'une des mesures phares des assises de la santé mentale qui ont été annoncées par le président de la République, hé bien c'est la prise en charge pour l'ensemble de la population dès l'âge de 3 ans, 2 séances chez le psychologue en ville, cette mesure doit permettre d'améliorer l'accès aux soins en santé mentale et s'adresse évidemment aux enfants et aux adolescents qui serait victime de harcèlement et pour toutes ces je vous demande le retrait de votre amendement, à défaut, j'y serai défavorable merci. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse de la commission. Et un avis d'une demande de retrait du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent, l'amendement est adopté. Un amendement 27 madame brûle. que demander de rapport dans 2 amendements successifs cette un peu trop pour le Sénat, et j'en suis désolé mais pour être tout à fait transparente, je ne pouvais pas rater l'occasion, et nous ne pouvions pas raté l'occasion puisque nous en sommes un certain nombre à plaider en ce sens de dire que si nous voulons vraiment être opérant face au harcèlement, alors il faut des moyens pour la santé scolaire, il faut des moyens pour la médecine scolaire qui se dégrade et dont les effectifs se dégrade de manière très alarmante, ne le voit, particulièrement dans le contexte de crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, où en gros des mesures que je qualifierais de bon sens et d'intérêt général qui aurait commandé qu'on puisse tester les enfants par exemple à l'école ne peuvent pas l'être, tout simplement parce que notre santé scolaire être indigente aujourd'hui et donc on ne peut pas identifier des fléaux des phénomènes d'une nouvelle nature comme celui dont nous débattons aujourd'hui avec tout ce qui a été dit sur le cyber-harcèlement etc qui fait prendre un tour nouveau au phénomène de harcèlement scolaire. On ne peut pas, comme vous venez de le dire, Madame la Ministre, montrez en quoi la santé psychique est un véritable enjeu pour les jeunes et les enfants, et encore une fois, dans le contexte que nous vivons et ne pas prendre 2 minutes comme je viens de le faire pour plaider en faveur de véritables moyens alors c'est pas une question simple puisqu'on manque de médecins globalement dans le pays et donc a fortiori dans la médecine scolaire, mais je crois qu'il faut engager un très grand effort de formation dans ce pays il y a une appétence pour les jeunes à s'engager dans les études d'infirmier dans les études de médecine, je crois que c'est le moment ou jamais d'engager cette. Faure, je vous remercie, C'est un avis défavorable, Céline Brulin s'y attendait, parce que d'abord c'est effectivement pas la tradition du Sénat mais surtout parce qu'on n'a pas besoin d'un rapport pour savoir que les moyens de la médecine scolaire sont insuffisants, alors le le plaidoyer de Madame Brunet a été brillant mais je pense que le rapport est est inutile. Avis défavorable. l'avis du gouvernement. Je ne mets effectivement que le plaidoyer était vibrant mais permettez-moi tout d'abord, Madame la sénatrice Brulin, vous me donnez l'occasion au travers de cet amendement de de rappeler sur le fond, combien le rôle des médecins, des psychologues, des, des, des infirmiers scolaires est essentiel dans la politique de lutte contre le harcèlement scolaire et combien leur accompagnement aux élèves est important et je tiens ici devant vous, à les en remercier toutefois et vous ne serez pas surprise, ce sujet a fait l'objet depuis 2006, d'une vingtaine de rapports déjà qui ont émané d'organismes de contrôle, tels que les inspections générales, les cours des comptes et ou d'autres assemblées d'experts et nous pensons qu'un rapport supplémentaire ne ne seraient pas très utiles, notre avis est donc défavorable. J'ai 2 demandes d'explications de vote monsieur fille merci monsieur le président, moi non plus je ne suis pas spécialement favorable à un grand nombre de de rapport, mais plutôt une action, je voudrais simplement profiter finalement pour peut-être qu'on recentre un petit peu bien le le vocabulaire, on a, il faut qu'on parle davantage de santé scolaire que de médecine scolaire, ce n'est pas une maladie, la la scolarité et la la 2ème chose le bien-être, la santé, c'est le bien-être physique, psychique et social des individus et si on qu'on sait quel est le le l'État démographique des des médecins, donc il faudra des années maintenant pour pouvoir combler tous les retards du numerus clausus, on sait aussi quelles sont les les besoins en infirmiers, infirmières des des services des même des services à domicile, en revanche on peut beaucoup plus facilement trouver des psychologues et on voit bien dans la santé scolaire, ce qui est souvent important, c'est justement le recrutement des psychologues faut d'ailleurs moins de temps pour pour former, c'est-à-dire qu'on peut engager une en rattrapage beaucoup plus important et en plus il y en a sur le marché, qui peuvent être à temps complet ou à temps partiel affectée, justement, à la santé scolaire dont le rapport sur le harcèlement prouve bien que c'est important. Monsieur dessus. Merci monsieur le président, a effectivement un rapport, on n'en a pas encore de les chiffres, on les connais, je les ai énoncées dans ma discussion générale mais il y en a un qui est écrit en c'est moins 15 % de médecins scolaires en 5 ans, on peut dans la durée du mandat donc c'est c'est quand même assez flagrant et là, c'est là qu'on regrette l'absence de du ministre Blanquer sur le banc aujourd'hui parce que ça nous aurait permis de débattre de ce sujet puisqu'il y a quelques semaines, on n'a pas pu débattent du budget de l'Éducation nationale et de ces questions-là, donc on aurait bien aimé en débattre aujourd'hui on aurait bien aimé débattre parce que c'est le le harcèlement scolaire c'est aussi un ça aura aussi un grand débat sur la santé mentale des adolescents.

pour rester ouvertes, notamment en terme de, de, de, de santé lors de santé scolaire puisqu'il faut utiliser ce terme désormais donc je soutiendrai cet amendement. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Quels sont ceux qui sont pour. Qui sont contre. Qui s'abstiennent. L'amendement n'est pas adopté.

Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues par cet amendement, nous souhaitons que les conseils d'école et d'administration des établissements puissent au moins une fois par an, bénéficier d'une information de la part des associations de lutte contre le harcèlement scolaire et du chef d'établissement sur la coopération existant entre ces associations et l'établissement et qu'un débat puisse avoir lieu, l'Assemblée nationale avait prévu un dispositif permettant de renforcer les Liens entre les établissements d'enseignement scolaire et ces associations de lutte contre le harcèlement scolaire et le soutien aux victimes, ça aide rédaction place et et place dans et la place dans le code de l'éducation n'était pas idéale, nous préférons donc lui substituer un dispositif donnant aux organes exécutifs des établissements les moyens de débattre de la politique de mise en oeuvre et à envisager, avec le soutien des associations compétentes de mieux lutter et mieux prendre en charge le fléau que constitue le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, ces associations sont très actives et demandeuse de davantage de Liens avec les écoles et établissements scolaires il serait positif qu'un plan d'action pour la prévention et pour la lutte contre le harcèlement, ainsi que pour la prise en charge de ces victimes de ses auteurs et de ses témoins puissent être débattue et arrêté annuellement par les conseils exécutifs des établissements, je vous remercie. Monsieur le président, Madame Voynet, je donnerai un avis défavorable, malheureusement sur cet amendement pour 2 raisons : le 1er raison relative au fait que, ou vous évoquez les, les, les conseils d'école, mais dans le secondaire, ce sont les conseils d'administration qui seront concernés, or ce n'est pas le l'instance la plus appropriée pour évoquer la problématique du harcèlement scolaire, celle qui est la plus appropriée, c'est ce qu'on appelle maintenant le comité d'éducation à la citoyenneté, à la santé et à l'environnement. Il me semble, il ne faut pas charger encore les conseils d'administration, la 2ème raison, elle est liée au caractère obligatoire que vous souhaitez donc instauré dans le partenariat avec les associations, les associations, alors je pense à Marion, la main tendue à Hugo font un travail formidable et beaucoup d'établissements scolaires saisissent le savoir-faire : l'expérience de ces acteurs associatifs pour les faire venir dans leur établissement pour faire des des séances de de prise de conscience, il y a des ateliers tout à fait formidables mais il ne faut pas obliger tous les établissements de France à agir ainsi. La liberté du chef d'établissement, la liberté des enseignants à agir, me semble une des bases de notre système éducatif et il faut rester dessus : avis défavorable. Monsieur le Président, peut-être juste pour revenir un instant sur la remarque de Monsieur le Sénateur, je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que Jean-Michel Blanquer, avait été retenu au Parlement européen ce matin et, manifestement, vraisemblablement, les débats vont se poursuivre cet après-midi et il devrait être à vos côtés, madame la sénatrice Egg. L'expertise et l'appui des associations spécialisées dans la lutte contre le harcèlement sont régulièrement sollicités par les établissements et elles interviennent auprès des élèves et des personnels pour des actions de sensibilisation et nous n'avons pas besoin de la loi pour permettre aux établissements scolaires de s'appuyer sur les associations dans la lutte contre le harcèlement scolaire, par ailleurs, un comité national d'experts a été créé en mai 2018 il est multi-elle t'elle est spécialisée dans les questions de harcèlement il. S'associe à des partenaires associatifs des inspections générales des experts universitaires, des médecins, des professionnels de terrain, des membres du ministère des influenceurs, des médecins, spécialistes des médias et il a pour rôle d'appuyer le ministère dans sa politique nationale de prévention. En faisant notamment du partage d'expertise et en étant un relais de l'éducation nationale sur le terrain, il y a eu des actions en cohérence avec le plan d'action du ministère de l'Éducation nationale, il y a des contributions écrites et des interventions dans les séminaires et dans les classes, il est de ces compétences également de favoriser le travail partenarial avec les associations et donc conformément à la vie, qui avait été donné par le gouvernement à l'Assemblée nationale, nous vous demandons le retrait de cet amendement, sinon ce serait un avis défavorable.

et notre collègue a beaucoup travaillé sur ce cette problématique du harcèlement scolaire par compte vraiment, je voudrais lui dire que je suis très attaché aussi à la liberté d'organisation, la liberté d'administration et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'inscrire cela dans la loi à un moment où on sollicite les associations ou ces associations ont ont eu beaucoup de mal pendant ces 2 années de pandémie si on rend obligatoire, il faudrait qu'on soit aussi assuré qu'il y aura suffisamment d'associations et de bénévoles pour pouvoir intervenir dans tous ces établissements voilà donc je suivrai l'avis du rapporteur.

il nous semble au contraire extrêmement important de rendre obligatoire pour tous les établissements, une telle coopération avec les associations en charge de la lutte contre le harcèlement scolaire et de prévoir un débat annuel dans leur conseil le phénomène de harcèlement produit trop de dégâts, souvent irrémédiable pour qu'aucun établissement ne puisse se dispenser de cette séance annuelle aucune école, aucun collège, aucun lycée n'est malheureusement à l'abri de la survenue de harcèlement en son sein le rapporteur nous indique par ailleurs qu'il relève de la compétence du comité à l'éducation à la citoyenneté, plutôt que de celle des CA de traiter de cette question, encore faudrait-il que ces instances soient réunies et régulièrement quand elles le sont, ce qui est loin d'être le cas dans de nombreux établissements, pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement. Merci. Je vais mettre aux voix, c'est cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission, une demande de retrait du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Ils s'abstiennent l'amendement n'est pas adopté l'article 3 bis restent supprimés. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 15 heures pour l'examen de la proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et à créer les instituts régionaux de formation, la séance est suspendue.